J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 n'est pas parvenu à l'adoption d'un texte commun. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d'élus, de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal un édile victime d'agressions, présenté par Madame Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues demande du groupe du Rassemblement démocratique et social européen dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la reporter, mes chers collègues. en 1er lieu évidemment remercier Nathalie Delattre et et son groupe pour cette proposition de loi, il est un peu regrettable qu'en 2022, il faille une loi pour protéger les élus, avouez que c'est quand même une situation un peu grave, ils ne sont plus à l'abri des violences les plus graves, le président Larché a l'habitude de dire les élus locaux et les mères sont à portée d'engueulade, les engueulades, certes, mais les violences physiques, les délits et etc, évidemment c'est tout à fait inacceptable, nous avons tous en tête la mort du maire de signes Jean Mathieu Michel, le 5 août 19 2019 qui avait entraîné d'ailleurs une une consultation de la part du président questeur et un rapport d'ailleurs qui a suivi, qui étaient extrêmement intéressant, alors évidemment nous sommes d'accord avec ce qu'a dit Madame Delattre tout à l'heure en en en

tentative d'étranglement d'homicide a lâches agressions avec couteau de cuisine, pris à partie et bousculé avec force contre un mur, agression avec fourche à 2 dents pointé sur le ventre, agressions physiques en mairie, coup de poing avec 4 jours d'ITT, c'est ce qui figure dans le rapport de de Philippe Bas pour être intervenu sur une nuisance sonore dit Lemaire, j'ai été agrippé par la personne qui voulait me casser la gueule, bref un automobiliste en contresens auquel j'ai indiqué son incivilités de coups de poing dans la figure, je veux dire, on est très très loin de de l'engueulade, des centaines de de pneus crevés, des voitures brûlées, des incendies de maisons des tags sur la maison des destructions de de clôture, bref, le rapport de Philippe Bas de 210 de 2019 est absolument effrayant cette triste réalité touche l'ensemble des territoires. Et les zones rurales ne font pas exception : la période de crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la situation et les derniers chiffres sont peu encourageants, les agressions physiques contre les élus ont augmenté de 47 % les 11 premiers mois de 2021 par rapport à la même personne, à la même période de

de classement sans suite d'une justice trop longue de sanctions qui n'était évidemment pas rendu ou alors très tardivement, vous allez vous avez devancé ma demande, parce que tout à l'heure, hé ben voilà, puisque tout à l'heure dans votre intervention, vous avez indiqué que vous aviez, par circulaire, donné des instructions et finalement répondu par avance aux questions que nous pouvions nous poser, donc très bien, vous m'avez évidemment retiré le le pain de la bouche de mon n'intervention il il revient maintenant évidemment au au parquet de faire le nécessaire dans ce sujet qui est un sujet éminemment important puisqu'on dit que les maires sont les élus préférés, il n'en reste pas moins vrai que le climat de violence qui sévit partout ne les épargne pas donc évidemment il est absolument nécessaire de voter la proposition de loi présentée par Madame De Lattre et par par son groupe qu'il convient encore une fois, de féliciter de remercier espérer que le cheminement vers l'Assemblée Nationale nous conduisent à un texte qui soit aussi adopté par l'Assemblée nationale, dans des délais relativement courts adoptée et dans des délais courts regretté que nous ne soyons pas aller plus loin en l'état, puisque l'élargissement proposée à l'article de 19 du code de procédure pénale ne permettra pas aux associations de contraindre le parquet a engagé des poursuites, mais si déjà vous non mais ça c'est pas possible, et poursuites soient évidemment améliorer, c'est déjà un pas très important, je note que la quasi-totalité des souhaits de Philippe Bas dans le rapport qu'il l'avait rendu à l'époque ont été satisfaits, c'est donc évidemment avec enthousiasme que le groupe de l'Union centriste votera cette excellente proposition de loi merci, cher collègue. Alors la parole est normalement Monsieur ravi mais il n'est pas là, donc je vais passer la parole. Ah monsieur Éric Gold pour le groupe RDS. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de commission, madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre, co-signé par tous les membres du RDSE et inscrite sur notre première espace réservé de l'année, entend s'attaquer une réalité malheureusement vécu par de plus en plus d'élus. Plus de 1000 agressions ont été recensées en 2021 contre des personnes titulaires de mandats électifs pour la majorité des maires et des adjoints, probablement par ceux qui sont en première ligne, la vitrine de notre République, au Sénat, chambre des territoires ce phénomène croissant et malheureusement bien connu, chacun d'entre nous peut citer le cas d'un élu, victime d'agressions et pour certains même, l'histoire et personnel et le traumatisme vivace dans mon département, je pense au maire de Lussas roué de coups le matin même de l'ouverture du congrès des maires par un d'automobilistes à qui il demandait de rouler moins vite, je pense aussi à la mère de Valpellets qu'il a reçu lors d'une cérémonie des menaces de mort pour une histoire de conflits de voisinage ou encore à 2 autres maires du département qui ont vu leur maison personnelle taguée d'insultes et menaces, mettant leur famille dans un état de stress et d'insécurité intolérable. Il n'y a pas un jour sans que celles et ceux sur qui repose le bon fonctionnement de nos institutions fassent l'objet d'une défiance qui s'exprime trop souvent par la violence, dans certaines communes, il n'est même plus rare que les membres des familles enfin aussi l'objet d'incivilité, menaces et violences, du simple fait d'être le conjoint ou la conjointe, le fils, la fille, le père ou la mère d'un élu, la mesure de la dégradation des conditions d'exercice des mandats semble avoir été prise, le constat est unanime et certaines dispositions ont même été adopté mais la réalité demeure inacceptable et appelle à des actions supplémentaires. La proposition de loi de Nathalie Delattre prévoit ainsi de répondre à une demande de l'association des maires de France qui souhaite étendre la possibilité déjà accordés à ces antennes départementales de se constituer partie civile au pénal pour se tenir avec son accord, un élu victimes d'agressions. Le Champ des infractions concernées sera également étendu pour mieux prendre en compte la diversité des situations vécues sur le terrain. Rappelons que d'après la consultation lancée par le Sénat en 2019 un faible nombre d'agressions, d'élus, fait l'objet d'une plainte et qu'un plus petit nombre encore fait l'objet d'une condamnation. Le monde accompagnement est un frein majeur soulevé par les élus, notamment dans les plus petites communes, les associations d'élus qui disposent de l'expertise de ressources nécessaires, semble en effet les mieux placés pour épauler ceux qui souhaitent porter plainte avec tous les avantages que la constitution de partie civile confère pour l'accès au dossier, le soutien global de la victime. Il semble donc justifié d'étendre cette possibilité qui donnera plus de poids aux procédures enclenchées qui permettra à l'AMF de recouvrer les sommes engagées pour la défense des élus agressés et qui incitera les autres associations d'élus, je l'espère, à mettre en place des accompagnements ciblés analogues. Faisons le constat que le service public s'apparente, pour une part croissante de la population à un simple biens de consommation courante, j'avais souhaité en 2019, renforcer la législation en déposant une proposition de loi visant à lutter contre les incivilités menaces et violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif local 100 déclinerait une partie à travers 3 amendements qui pourraient compléter les dispositions de cette proposition de loi, l'absence de réponse forte à ces situations augmentent évidemment le sentiment d'abandon et découragement des élus, notamment en zone rurale où la réponse est insuffisante en matière de constatation des infractions d'enquête de durée des procédures et des décisions. les débats et les propositions qui vont suivre, nous permettront, je l'espère, d'améliorer la situation pour ceux qui sont en attente légitime de réponse, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur André Richard. Pour le groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, ce le président de la commission madame la rapporteure, mes chers collègues comment commencer cette intervention sans remercier très chaleureusement notre collègue Nathalie Delattre pour avoir pris l'initiative de cette PPL texte ce texte et inscrit dans la compte continuité de diverses initiatives prises par le passé, et notamment par le Sénat qui ont considérablement renforcé la protection des élus en cas d'agression. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler que l'article de tirer 19 du code de procédure pénale dont la PPL propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 1er est issu d'un amendement sénatorial à la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, mais dans le contexte que l'on connaît d'augmentation des agressions contre les maires, et plus généralement des élus la PPL de Nathalie Delattre est venu judicieusement boucher les trous dans la raquette comme on dit, ainsi dans sa version initiale, d'une part, elle a élargi la possibilité de se porter civile en cas d'agression d'un élu local à 3 associations nationales représentant les différents niveaux de collectivités territoriales, l'AMF l'ADF et régions de France, mais d'autre part et surtout, selon moi L à RG, elle a élargi les motifs pour lesquels ces associations pourront désormais se porter partie civile ainsi au cas d'injure ou outrage, diffamation, menaces ou coups et blessures déjà visées par le code de procédure pénale s'ajouteront judicieusement les destruction, dégradation ou détérioration de biens et la divulgation d'informations dans le but de nuire à une personne exposant cette dernière a un risque en outre ces infractions seraient prises en compte, non plus seulement lorsqu'elles visent des élus investis d'une fonction exécutive, mais également lorsqu'elles concernent des membres de conseils municipaux ou de conseils départementaux et régionaux, elles pourront même visées non seulement l'élu lui-même, mais également un membre de sa famille lorsque c'est en fait l'élu qui est visé en raison de son mandat ou de sa fonction, on le voit, mes chers collègues, ces élargissements paraissait bienvenue car particulièrement circonscrit et cohérent, on aurait d'ailleurs pu s'en arrêter là, la commission des lois, monsieur le président, en a décidé autrement on enrichissant dans un 1er temps le texte par des amendements nos collègues Kader d'une part le rude, d'autre part, les premiers ont encore étendu les infractions au titre desquels la constitution de partie civile et pas est possible avec la prise en compte des actes d'intimidation et de harcèlement des violations de domicile et des atteintes volontaires à la vie l'amendement monsieur de rudes, a permis aux assemblées parlementaires et aux collectivités territoriales de se porter aussi partie civile en cas d'agression de leurs membres ou de leurs proches, désormais, peut-on dire les trous dans la raquette paraissent bel et bien remplie pour autant nous étions quelques-uns au sein de la commission des lois, se demander pourquoi cette possibilité se porter partie civile n'avait pas, n'avait été élargies qu'aux seuls 3 associations nationale, cité dans le texte, d'autres associations nationales ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des élus auraient également pu intervenir légitimement à cet égard, il n'y avait d'ailleurs aucun risque particulier à élargir de la sorte, dès lors qu'on le sait, aucune procédure ne peut être engagée sans l'accord de la victime et pas plus qu'avant le nouvel article de tirer 19 ne permettra aux associations de contraindre le parquet a engagé des poursuites en réunion de ce jour, avec l'accord de l'auteur de la PPL et après concertation avec le gouvernement, monsieur le garde des Sceaux, la commission a décidé de faire droit à cette sollicitation à cette sollicitation et propose un texte qui, à mon sens peut largement faire consensus dans cet hémicycle, il le fera assurément pour ma part je le voterai avec enthousiasme en saluant tout particulièrement la co-construction qui a précédé présidé à son élaboration, ce qui n'est pas un mes chers collègues, aussi banale que ça et qui illustre clairement l'attachement et particulièrement bien l'attachement d'user du du Sénat aux élus locaux, vous me permettrez, enfin, de formuler un dernier voeu, je souhaite que ce texte puisse contribuer à terme au moins un peu à réduire, voire 100 sanglier données supprimer les uns les intolérable agression d'élus dans ce pays, je vous remercie. la parole est à monsieur Joël Guerriau pour le groupe, les indépendants. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne peux m'empêcher à mon tour et à titre préliminaire de rappeler à cette tribune le dévouement à la sable des élus locaux et notamment des élus municipaux qui sont au service de nos concitoyens et qui assure le bon fonctionnement de nos territoires, synonyme d'écoute et de proximité, l'élu local en oeuvrant dans l'intérêt général, fait vibrer la démocratie au quotidien, il agit pour la République avec courage et loyauté. Or, depuis plusieurs années déjà, sur l'ensemble de notre territoire, nous constatons une multiplication des atteintes physiques ou verbales auxquelles les élus locaux sont confrontés dans l'exercice de leur mandat et je pense que le moindre fait doit être prise en considération pour illustrer mes propos, je pense en particulier à une affaire qui est récente dans notre département, un maire qui s'appelle Bruno Debray qui est, d'après qui est maire de sur les mines qui est une commune de moins de 2000 habitants, est interpellé par une habitante qui le signale un incident l'incident, c'est très simple, c'est qu'une dame qui se promène avec sa poussette et qui a un petit chien se trouve agressé par 2 de de gros chien qui agresse ce petit chien mais avec le risque bien évidemment de des conséquences assez dramatiques, heureusement, très vite, il y a une intervention, tout se passe plutôt bien, le maire, le lendemain, va voir la propriétaire et le signale les faits en lui demandant pour la suite, très poliment, de bien vouloir mettre ses chiens en laisse. Que n'a-t-il pas fait le mari furieuse se précipite à la mairie s'introduit dans le bureau du maire et l'insulte, la Grèce verbalement le maire bien évidemment porte plainte, mais l'affaire est jugée sans suite, quelques temps plus tard, nouveau fait qui est porté l'attention du maire, le fait que la coiffeuse c'est vu agresser parce que les enfants de cet individu aurait été mal coiffée, donc elle a été tenu de rembourser la coiffure mais que pouvait-il faire le maire de de désormais puisque manifestement, il se sent impuissant dans l'exercice de son mandat et le respect de son autorité, voilà que tous les faits sont importants, bien sûr, nous gardons tous ici en mémoire, comme l'a rappelé Nathalie a défait bien plus tragique, celui de signes en août 2019 le maire Jean Mathieu Michel a brutalement perdu la vie, renversé par une camionnette alors qu'il venait d'empêcher le dépôt de sauvages de gravats. Bien sûr qu'il y a des faits bien plus graves mais c'est tous les tout tout toutes ce qui peut toucher l'autorité du maire qui doit être traitée, face à la recrudescence de ces agissements d'individus défiant l'autorité de la puissance publique agissements que notre République ne saurait tolérer, nous devons et nous l'avons tous dit mieux soutenir les élus locaux, c'est pourquoi, à l'initiative de notre collègue Nathalie Delattre et bien sûr la bienvenue en donnant la possibilité aux différentes associations nationales d'élus de que se constituer partie civile pour accompagner au pénal tout édile qui aurait donné préalablement son accord lorsqu'il est victime d'agressions et de harcèlement, nous aussi, en cas d'infraction d'Exposition délibéré un risque grave par révélation d'informations privées ou encore en cas de dégradation d'un de ses biens ou enfin lorsque la victime est l'une et l'un de ses proches, nous avons si un cas en Loire-Atlantique ma collègue qui était si présente connaît aussi bien que moi ce cas c'est une femme qui est maire de vue étaient régulièrement harcelés au conseil municipal par l'ancien maire, ce qui peut vous dans le public, est ce qui est une affaire qu'on n'arrive pas à régler cette initiative est également pertinente cette loi parce que à la tâche à mon sa tâche à mentionner expressément que les associations d'élus peuvent accompagner tous les élus victimes, même ceux qui ne sont pas investis de fonctions des apports importants ont été ont permis d'enrichir la proposition de loi lors de son examen en commission, je me réjouis donc ainsi que la liste des infractions au titre desquels la constitution de partie civile est possible et puis être élargi aux actes d'intimidation de harcèlement de violation de domicile ainsi qu'aux atteintes volontaires à la vie, avec l'accord de en droit de la victime, nous nous fait si les si les citons également de la possibilité qui a été donné aux assemblées parlementaires et aux collectivités territoriales de se porter partie civile en cas d'agression d'un de leurs membres ou de leurs proches

Madame la présidente, monsieur le Ministre. Madame l'auteur merci madame De Lattre pour cette proposition, madame la rapporteure, chers collègues, il n'aura échappé à personne que notre société se polarise que les tensions sont exacerbées et que les élus, mais pas que font l'objet souvent du de colère mal placé des violences jamais justifié sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, publié en janvier 2021, ils ont déjà été cité des violences physiques entre les élus ont augmenté de 47 % sur les 11 premiers mois de 2021. Dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints

mais encore une fois, ni la frustration de la compréhension des décisions personnelles ni la fatigue, parfois devant la complexité et la lenteur de certaines administrations ne saurait justifier de quelconque violence, elle est toujours justifiable la violence dans ce cas à l'égard des élus de leur pays, plus de 300 plaintes pour menaces de mort, a été déposée et plusieurs sources rapportent une hausse de ces violences, ces élus qui caustique, il continue malgré les difficultés, c'est un euphémisme, à se mettre au service des autres méritent une protection et les récents textes ont déjà accru cette protection la présente proposition de loi s'inscrit dans cette démarche, tant mieux mais permettez-moi quelques réflexions, malgré tout, ce n'est pas le 1er texte qu'il m'ait permis de discuter au nom de mon groupe qui m'interroge sur la volonté du d'ultra spécialisation des textes selon les victimes, il est peut être Live de ma part d'importantes de répéter l'égalité de la loi et la perception de l'égalité devant la loi et le fondement de notre société démocratique je ne reviens pas sur le vous êtes condamné les agressions de matières spécifiques pour les représentants des citoyens, les représentants de l'État et personne chargée d'une mission de service public, mais j'aurais du mal à justifier auprès de mes concitoyens et même de nos électeurs pourquoi l'agression de leur famille, devrait connaître une sanction plus sévère que l'agression de la famille, de ses concitoyens.

l'amendement déposé par la rapporteuse de la commission des lois, dont on a parlé, ne me semble pas spécialement arranger les choses, en ajoutant la notion de personne vivant habituellement à son domicile. Je prends un exemple mais se cuise de le prendre plus trivialement mais la nounou de la concubine du neveu hébergé par exemple, le jardinier à demeure de la belle-mère du concubin de sa fille abrités sous le même toit, peut-être pour la circonstance, je peux citer d'autres exemples je sais bien que la loi n'est pas fait pour ça, mais malgré tout, il faut quand même essayer de voir où nous pourrions en arriver avec ce type d'abonnement, nous comprenons et entendant le sentiment de lassitude des élus agressés, je rencontre autant que vous tous les jours et il demande plus de sévérité, même si la solution ne se trouve pas forcément dans l'aggravation des délits sanctionnés de manière plus importante ou l'extension d'une plus grande protection aux personnes relevant de la sphère privée des élus la suffisance des moyens humains et matériels de la justice et souvent responsable de sa lenteur et elle reste structurelle et profonde et demande encore une croissance substantielle du budget de la justice dans l'objectif d'augmenter le nombre de magistrats et de greffiers et de greffiers pour pallier ces dysfonctionnements pour autant nous accueillons favorablement l'idée d'élargir la protection à l'ensemble des élus, il est aussi essentiel de mieux accompagner les élus et nous partageons la pertinence de la constitution comme partie civile, des associations d'élus, leur intérêt déjà reconnu au niveau de leur filiale locale, il apparaît opportun de l'élargir aux associations nationales, nous porterons 2 amendements là afin de prendre en compte les outrages sexistes, l'autre car nous souhaitons élargir la possibilité de se constituer partie civile au delà des grandes associations nationales comme l'Association des maires de France, c'est un désir partagé par un grand nombre d'entre vous, puisqu'il y a de nombreux amendements déposés à ce sujet, l'idée d'un monopole d'accompagnement de la terre et agir nous paraît problématique juger la qualité de l'AMF voilà chers collègues dans sentiment profond aux inquiétudes réelles sur un sujet essentiel, mais dans tout débordement s'apparentant à une volonté de justice corporatiste serait nuisible et contre-productive dans l'ambition d'une meilleure protection des élus.

Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, c'est le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, dont l'auteur de la proposition de l'Nathalie Delattre à septembre 2021, l'hôtel de ville de Kongou dans mon département, a été la cible d'un incendie volontaire après des manifestations contre la destruction d'un bidonville un mois plus tard, les véhicules du maire de Ouaga ni de sa femme et d'un autre élu de la municipalité ont connu le même sort, plus récemment, le maire de Bandrélé a fait l'objet de plusieurs menaces de mort, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, publié en janvier 2022 plus de 1100 élu majoritairement des maires ou leurs adjoints ont subi des agressions et 400 outrage ont été recensés lors du congrès de l'AMF de novembre 2021, le président de la République, rappeler la nécessité d'être intraitable face au retour et à l'augmentation de la violence envers les élus et particulièrement les mères dépositaires de l'autorité publique, le chef de l'État avait estimé que la sanction devait être décisive par devoir envers nos élus, la proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans cet état d'esprit en apportant une réponse à une demande de l'AMF de se porter partie civile lors d'agressions, d'élus, initialement composé d'un article unique, elle a été enrichi lors de l'examen par notre commission des lois, ainsi les principales associations nationales d'élus AMF AMRF ADF et régions de France pourront se constituer partie civile pour accompagner au pénal : tout est dit-il de l'hexagone et des outre-mer qui aurait donné préalablement son accord, notamment en cas de dégradation d'un de ses biens d'agression d'actes d'intimidation de harcèlement et de violation de domicile, leurs proches pourront également en bénéficier, je me permets de saluer la rédaction de compromis trouvé sur l'article 1er entre notre rapporteur et le gouvernement, en outre, la divulgation d'informations dans les, dans le but de nuire à une personne adopté dans le cadre de la loi, confortant le respect de principes de la République constituera elle aussi une infraction les assemblées parlementaires, les collectivités territoriales et le Parlement européen auront la possibilité de se porter partie civile en cas d'agression d'un de leurs membres ou de de ses proches, enfin et grâce au travail réalisé par notre rapporteur, ce texte s'appliquera en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna viendra étouffer les actions d'ores et déjà menées par le gouvernement et notamment le ministère de la justice avec la direction des affaires criminelles et des grâces, ainsi que le ministère chargé des collectivités territoriales, je pense à la circulaire du 7 septembre 2020 adressé au parquet, mettant en oeuvre une politique pénale ferme ou encore celles du 15 déc 2020 relatives à la mise en oeuvre de la justice de proximité pénale pour une justice plus proche des partenaires locaux, je pense également à l'article 34 de la loi Engagement et proximité qui est venue renforcer la protection juridique et la formation des élus locaux face aux violences et aux incivilités, enfin je salue l'initiative du Sénat, de mettre en place une formation organisée par la DGPN, sur la sensibilisation des sénateurs à la gestion des comportements agressifs et à la désescalade du conflit, tant que vigie des territoires, nous pourrons grâce à cela, accompagné et aidé nos élus face aux agressions, les élus de la République doivent être protégé dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur vie privée, les accompagner et renforcer la réponse pénale, c'est pourquoi le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de loi. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure madame l'auteur de la loi cette proposition. Pour objectif, nous l'avons dit redit depuis le début de cette séance de soutenir les élus dans leur démarche judiciaire des marches qui peuvent engager la suite notamment de violences commises à leur encontre, elle permet aux associations d'élus, de les accompagner dans ses démarches au pénal, on ne peut que saluer cette initiative portée par notre collègue présidente Delattre, car les élus sont très régulièrement la cible d'attaques dans la violence intitule s'intensifie d'année en année je pense bien sûr aux maires d'abord Homer qui semble être au centre de nombreuses revendications de leurs concitoyens et qui représentent la grande majorité des victimes bien sûr plus entre vous l'ont cité le c'est terrible, presque assassinat en tout cas, en tout cas, homicide volontaire sur le maire de signes mortellement renversé que nous ce qui nous a tous tes tous marqués la violence dans les élus municipaux font l'objet peut s'expliquer par leur rôle de 1er plan dans la vie des Français, ils exercent des responsabilités, prennent des décisions pas toujours populaires qui impacte directement le quotidien de leurs administrés et leur visibilité les rend facilement identifiables à portée de baffe, ça vient d'être dit, dès lors, il cristallise les critiques, les revendications et dans les cas les plus graves, peuvent faire l'objet d'agressions ces actes, nous devons les condamnés tous sans exception, car la violence n'est jamais la solution pour cela, la justice doit être saisie, mais ils ont besoin de soutien, de moyens de ressources, certaines associations d'élus possède ses ressources et peuvent apporter un accompagnement bienvenue en pareille circonstance, et tout l'esprit de la loi, la rédaction initiale de cette proposition prévoyait que seul l'AMF l'ADF, l'ARF pouvait se constituer partie civile je reconnais évidemment le travail de ces 3 grandes associations ces majors en tant que telle, cependant, il me semble que chaque élu doit pouvoir se faire représenter par l'association qu'il juge la plus adaptée pour défendre ses intérêts, j'avais donc déposé un amendement en commission pour elle : élargir le Champ des associations à toutes celles qui le prévoit et qui sont régulièrement enregistrés cet amendement avait été madame la rapporteure rejeté en commission, il faut jamais avoir raison trop tôt, manifestement, heureusement et je m'en réjouis, il semble qu'une semaine plus tard avec la réflexion est telle ou telle intervention, le gouvernement étant entendu notre appel et a souhaité que la rapporteure, dépose un amendement qui va dans le même sens, nous verrons cela tout à l'heure et c'est tant mieux, le Champ des infractions visées de être plus large possible, car nos élus sont la cible d'attaques physiques contre leurs biens ou leur encontre mais aussi l'attaque verbale, c'est aussi un amendement qui a été intégrée dans par la Commission dans le Champ de la PPL, je m'en réjouis, mes chers collègues, je voudrais revenir sur un point : l'actualité qui vous a tous je crois marqué pour ne pas dire choqué l'exemple de Louis Boyard. Député de la France insoumise. Insulté par Cyril Hanouna et le dernier exemple en date, oh combien révélateur de ce que nous évoquons aujourd'hui et qu'on peut résumer sous le vocable de vulgarisation de notre audiovisuel l'escalade d'absurdité de violence à laquelle nous avons assisté lors de cette séquence télévisuelle n'a existé que pour répondre à cette soif de petites phrases qui fait le Buzz, ce qui n'est digne ni de la classe politique, ni de la classe journalistique, je ne peux que regretter, je ne peux que regretter que tout soit érigée en polémique pour que l'on en parle à ce petit jeu, les gagnants sont toujours les mêmes, ce sont les extrêmes et il nous appartient en tant que politique, de ne pas se prêter à ces petits jeux. Notre discussion du jour porte sur une proposition d'amélioration de l'accompagnement des élus lorsqu'il décide d'engager des poursuites contre les auteurs d'agressions, on ne peut qu'y souscrire d'ailleurs le calendrier nous y invite, d'autant plus à une semaine du congrès des maires, quelle belle opportunité, les élus locaux jouent un rôle majeur dans notre pays, ils sont plus de 500000 à exercer un mandat local à nous représenter à nous défendre, a défendent l'intérêt général à travers élaboration à la mise en oeuvre de politiques publiques lorsqu'on leur donne les moyens et je fais ici une parenthèse qui devrait nous réunir, très largement, à savoir que, aujourd'hui, ces moyens sont de plus en plus fragilisé les maires sont fragilisés dans l'exercice de leur mandat, car on leur demande toujours plus avec des moyens de plus en plus limités, ils sont inquiets de l'augmentation de leurs charges, ils sont inquiets que c'est Charles ne suivent pas le niveau de l'inflation, ils sont inquiets que les dotations puisse être potentiellement diminuer bientôt dans le cadre du PLF, mes chers collègues, nous saurons je crois répondre à leur légitime inquiétude, il faut des recettes pour permettre au budget d'investissement obligé de fonctionnement d'exister et surtout de mettre en place les projets, souhaitée par nos concitoyens, tout cela participe à une fragilisation de l'image de l'élu, quand il ne peut pas agir bien évidemment et je le dis à un membre du gouvernement, aujourd'hui il y a une grande inquiétude qui s'exprimera aussi à l'occasion du congrès des maires, mes chers collègues, pour conclure cette action des élus locaux irriguent l'ensemble de notre vie quotidienne, elle doit être respectée sans élu, il n'y a pas d'organisation de notre société possible, il est évident qu'en cas de violence, il faut mettre à leur disposition toutes les ressources qui pourraient les aider dans la défense de leur intérêt et vous l'aurez compris mon groupe votera cette proposition de loi enrichis par les débats qui vont suivre, je vous en remercie. Merci monsieur le président, la parole est à madame Cécile. Sherman pour le groupe CRCE. Madame la présidente, madame la miss Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues, la PPL qui nous est présenté ce soir en temps effectivement permettre aux différentes associations la semaine nationale d'élus, de se constituer partie civile pour accompagner au pénal tout est dit-il, qui aurait donné préalablement son accord, les élus et, plus spécifiquement, les élus locaux sont les premiers contacts de nos concitoyens, avec l'autorité publique aujourd'hui l'article de tirer 19 du code de procédure pénale n'autorise l'action des associations qu'en cas de faits commis contre l'élu, à raison de ses fonctions particulières et non de son mandat, la PPL que nous examinons et donc utile égalitaire, en effet, grâce à son apport, elle envisage que les à sensation d'élus puisse accompagner tous les élus, victime de harcèlement ou d'agressions, même ceux qui ne sont pas investis de fonctions particulières et c'est en cela que nous la considérons pertinente, néanmoins, nous ne pouvons ignorer que le climat politique, économique et sociale actuelle étendu notre société va mal et de plus en plus d'hommes et de femmes sont inquiets et en colère contre les responsables politiques dans ce contexte, nous ne pouvons faire l'autruche, un élu incarnent des idées, des prises de position des revendications et nous sommes dans une démocratie et donc tout à fait sain de ne pas faire l'unanimité pour autant cette nécessaire opposition dans le débat d'idées ne doit pas justifier une attaque personnelle, physique ou verbale, et c'est bien parce qu'un mandat expose personnellement élu que cette PPL et comme je l'ai déjà dit à notre sens objectif la la qualité d'élu et depuis longtemps une circonstance aggravante pour plusieurs infractions, il convient également de se soucier de l'accompagnement des élus victimes tout au long d'une procédure devant le juge pénal cet accompagnement ne sera pas exorbitant de droit commun, étant donné que nos citoyens victimes peuvent également être soutenus dans leur procédure pénale par des associations à but non lucratif, il est donc adéquate pour répondre à cette attente d'accompagnement, d'étendre le Champ des associations susceptibles de se constituer partie civile, au-delà du soutien à l'élu lui-même : nous considérons qu'une telle action participe à la lutte en faveur d'un exercice serein des mandats locaux et donc du bon fonctionnement de nos assemblées locales un élu ne doit pas craindre pour sa personne dans l'exercice de son mandat et le risque d'une agression ne doit pas être dissuasif dans l'expression des opinions politiques, sauf à vouloir tuer la démocratie dans son existence la plus profonde aujourd'hui en droit pénal général, le fait qu'une personne chargée d'une mission de service public qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de sa mission est victime d'une infraction constitue une circonstance aggravante pour la majorité des infractions contre les personnes, cette aggravation des peines permet une réponse pénale satisfaisante en cas d'agression, mais aujourd'hui, le propos n'est pas celui de l'efficacité de la justice, mais celui de l'accompagnement de l'élu, un élu qui en tant que personne peut être traumatisé à la suite d'une agression, or aucun citoyen ne trois être isolé dans une procédure pénale qui pourrait le dépasser l'enjeu donc sous-jacent est celui de garantir le droit des élus à la liberté d'expression, nous ne devons craindre en raison de nos mandats le débat politique ne doit pas être vecteur de violence, l'art du débat doit être respecté en toute décence ainsi, nous considérons que la constitution de partie civile, des associations d'élus pour soutenir pleinement au pénal un édile victime d'agression est utile à un exercice serein des mandats électoraux et de la démocratie et, par conséquent, nous voterons pour cette proposition de loi, je vous remercie. la parole est à monsieur Jean Baptiste. De blanc pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, cher François Noël madame la rapporteure madame Di Folco, mes chers collègues, on propose 3 redondants, mais ça va mieux en le martelant la proposition de loi notre collègue Nathalie Delattre Perquis visant à permettre aux différentes associations d'élus, de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal un édile, victime d'une agression a été inscrite à l'heure du jour et c'est heureux, et même très heureux à travers cette inscription à l'Ordre du jour, nous voulons tous ici redire notre mobilisation sur le sujet, en effet, représentants des élus que que nous sommes, nous sommes tous les témoins des violences qui peuvent subir au quotidien, les maires et les élus de nos territoires,

la liste pourrait être beaucoup plus exhaustive, aujourd'hui, les agressions sont en effet d'une violence inouïe, injures, menaces de mort, agressions physiques, elles sont de plus en plus fréquentes touchent l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille et l'ensemble du territoire ce de manière physique et on le dira peut-être pas assez sur les réseaux sociaux aussi, où on se fait agresser et où on on se fait agresser, bien souvent de faux profils parfois, qui viennent de l'étranger, on pourrait aussi parler véritablement de cyber harcèlement des élus et qu'il faudra véritablement envisagé alors le rapport d'autres questeurs, Philippe Bas, dès 2019 avait très bien mis en lumière tout cela et c'est pour cela que les élus nous attendent tous pour des actes forts et immédiat, si l'on souhaite qu'il y a encore des candidats aux prochaines élections municipales forcé de constater que le dépôt de plainte, suite à la suite d'une agression est loin d'être systématique et particulièrement dans les petites communes

que la plainte sera rarement suivies d'effet, a tendance à prédominer alors trop souvent encore les maires et les élus se sentent seuls, face à ça, cette agression préfère se taire et faire comme si cela n'était jamais arrivé pour oublier le trimestre le traumatise, or nous sommes tous ici collectivement convaincus qu'il ne faut rien ne s'est passé, et que le dépôt de plainte doit être systématique et que nos édiles corvéables à merci dans leur commune mérité d'être mieux soutenus dans l'engagement d'une procédure pénale pour que justice leur soit rendue et les associations d'élus, y compris rural semblent être les mieux placés pour apporter ce soutien, par conséquent, l'adoption de cette proposition permettant aux différentes associations se constituer partie civile, sera un signe fort envoyé à tous les élus de ce territoire, nous avons, nous avançons donc tous petit à petit, vous-même, Monsieur le Ministre publié des circulaires, vous l'avez évoqué, invitant les parquets à mettre en oeuvre une politique pénale ferme et diligente répression des actes commis à l'encontre des élus locaux, ainsi qu'un suivi judiciaire, renforcer des procédures pénales et concernant, il faudra aussi que les juges s'approprient tous ces textes intériorise tous ces textes et s'habitue à avoir des élus dans les salles d'audience

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues. à portée de baffe, voici les mots qui me répète souvent mon maire Jean Léonetti au sujet des élus si j'ai souhaité intervenir sur ce sujet, comme vous tous ici présents, c'est pour dire tout haut ce que certains nous avoue tout bas pour cette année 2022 956 élus ont été pris pour cible en France entre le 1er janvier le 9 mai 956 en moins de six mois combien seront-ils donc à la fin de l'année, des chiffres en tout cas en nette augmentation, puisqu'ils sont déjà aussi important que pour l'année 2021 une année qui d'ailleurs enregistré déjà une hausse de 40 % de violence envers les élus par rapport à 2020 une époque : faut-il vraiment le rappeler ou nos collectivités territoriales et nos élus les locaux étaient plus que jamais mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire et pourtant, paradoxalement, ce n'est pas moins de 80 % des victimes, qui sont des élus municipaux, des chiffres qui invite à la réflexion, puisque les maires restent les élus en qui les Français ont le plus confiance, la proximité physique ne doit pas donc ouvrir un quelconque droit à la violence gratuite chaque intimidation vise en tout état de cause, à ce que les élus ne se sentent plus libres d'agir en leur âme et conscience, ces chiffres doivent nous alerter collectivement nous, parlementaires et gouvernement, mais avant tout, tous les Français la forte recrudescence de la violence envers les édiles est acté, obligeant l'Association des maires de France, d'ailleurs, a créé en octobre 2020, un observatoire des agressions envers eux, mais ce qui est plus alarmant, c'est que l'AMF a formé récemment 15000 maires et adjoints avec des formateurs du GIGN pour gérer les menaces et les situations de crise, je crois que quand un maire reçoit une formation du GIGN ou du Raid, cela veut dire quelque chose que le pays ne va pas très bien l'excellent rapport d'information de mon collègue Philippe Bas sur ce sujet, mettait d'ores et déjà cette triste réalité en lumière un faible niveau de plaintes associé un très faible niveau de condamnation, une violence qui progressent plus globalement vers l'ensemble des détenteurs de l'autorité en France ce dénigrement de l'autorité est au demeurant très très inquiétant : l'abstention électorale étant l'une des Mestre, manifestation à mon sens de cette crise civique des plus criantes, difficile à comprendre, en tout cas, impossible à tolérer, c'est certain, pire encore, c'est souvent par pudeur, mais aussi par peur de voir les menaces intensifier que certains élus préfèrent se taire se taire sur le fait de leur Perm que leur permanence a une nouvelle fois été vandalisée se taire sur l'énième insultes reçues en pleine rue, se taire sur la violence graduelle de ce qu'il sert au quotidien se taire alors pour ne pas déranger pour ne pas être pointés du doigt, stigmatisés, un drame est toujours possible, nous le savons, alors ne ben non, ils ont pas ces incivilités qui peuvent conduire au pire, c'est pourquoi je soutiens ce texte défendu par notre collègue Nathalie Delattre qui entend permettent donc aux différentes associations d'élus, de se constituer partie civile pour accompagner au pénal : tout est dit-il, qui aurait donné préalablement son accord, enrichi par le travail de la commission des Lois il répond aux attentes des élus victime de harcèlement ou d'agression qui mérite d'être mieux soutenus pour que justice leur soit rendue, je vous remercie. Merci, cher collègue, la discussion générale est Close. Nous passons à la discussion du texte de la commission et à l'article 1er 15 amendement faisant l'objet d'une discussion commune. En commençant par l'amendement 19 présenté par Madame Di Folco madame la rapporteure. Merci madame la présidente, alors oui, donc je vous propose par cet amendement une rédaction, une nouvelle rédaction de l'article 1er de cette proposition de loi je voulais indiquer, lors de la discussion générale, il est du sud. Du dialogue que nous avons menée avec le gouvernement, cette nouvelle rédaction tend à permettre à toutes les associations d'élus bénéficiant d'une ancienneté suffisante de se porter partie civile, tout en reconnaissant le rôle et l'implication de l'association des maires de France dans la défense des élus municipaux, c'est peut-être là que je vais un peu divergés par rapport à Monsieur le Président, Kader, c'était pas tout à fait perceptibles président ghanéen dans votre amendement, puisque vous faisiez fi de de l'AMF face à ce moment-là, cette rédaction paraît cohérente justement avec l'intention de l'auteur de la proposition de la loi et c'est vraiment ce qui comptait aussi, pour moi le bien respecter l'esprit initial de cette proposition et ça respecte aussi l'intention des auteurs, des amendements adoptés en commission sur cet article, hein. Et donc je vous sais. que par rapport au travail de la commission, nous avons accepté d'inclure le Parlement européen, ce qui n'était pas le cas où toute la semaine dernière, parmi les assemblées susceptibles de se porter partie civile Quentin de longuement mais agressé en ce qui concerne le Parlement européen, donc il s'agira des députés français et des députés étrangers lorsqu'ils sont victimes en France. Merci madame la rapporteure et nous avons un amendement identique numéro 23 à l'amendement Madame la rapporteure, présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci. La présidente je ne surprendrai personne en disant que je suis évidemment. Totalement en phase avec vous madame la rapporteure ces amendements qui sont identiques,

Sans remettre en cause évidemment ce qu'elle représente pour beaucoup d'élus, personne n'a évidemment l'intention de malmener l'AMF mais ne pas considérer les autres associations, c'était un vrai risque, quand un autre. Constitution cet amendement a par ailleurs notre mérite je dis mérite pardon c'est d'harmoniser et d'étendre le Champ des infractions dont les élus sont victimes. Voilà sommairement présenté cet amendement que nous avons madame la rapporteure en commun. Merci, monsieur le Ministre, nous passons à la présentation de l'amendement numéro 4 par Monsieur le Président, Kader. Oui, nous présenterons des amendements, madame la présidente, sachant que la l'adoption potentiel de l'amendement dix-neuf faire tomber tous les autres, bien évidemment, on est, a bien compris la la démarche qui a été engagé mais qui va malgré la remarque de la rapporteure qui va dans notre sens, c'est vrai que l'amendement que j'ai pu porter au nom de mon groupe ne mentionnait aucune association, estimant que les associations du Mans constatée ayant plus de 5 années de d'existence pouvaient légitimement revendiquer cette cette possibilité de défendre leurs élus, quels qu'ils soient donc voilà l'AMF l'ADF et l'ARF sont encore mentionné dans l'amendement de de la rapporteure, sans mentionner les autres associations très honnêtement, nous pensions qu'il aurait été plus simple de dire par là, toutes les associations d'élus, je ne sais bien que c'est pas tout à fait le sens qui était initialement pensé par madame De Lattre mais la simplification aurait permis d'éviter toute forme de concurrence entre le les secteurs associatif auquel nous allons de fait contribué, même si nous adopterons l'amendement dans la me dit Folco qui nous semble aller dans le sens fondamental sur lequel nous voulions amener la commission des lois, au moment où nous avons présenté ce texte, je vous remercie.

Oui, merci madame, madame la présidente, plusieurs intervenants ont évoqué parmi l'ensemble des maires qui sont victimes de ces agressions, les les maires ruraux et cet amendement visait à permettre à l'association des maires ruraux de France qui aujourd'hui représentative de de ces maires ruraux de pouvoir se constituer partie civile mais évidemment je me rangerai à l'amendement qui a été proposé, qui est élargie élargi cette possibilité à d'autres associations d'élus.

Il est identique, défendu.

Donc je me range un amendement qui est pris Je vais le défendre, enfin j'ai pas d'effort mais parce que c'est le même que ceux qui viennent d'être présentés, donc je défends quand même tous ces amendements là par rapport à ce qui a été présenté par le gouvernement et Mahdavi Folco pour point précis, je l'ai dit dans ma des discussions générales mais je le rappelle, le point précis c'est qu'il en est de même lorsque ces infractions sont commises, je passe sur le début sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, je trouve que cette notion-là et à la fois vague floue et peut donner lieu à de nombreuses exagérations voire, voire à de nombreuses manipulations, donc il n'y aurait pas cette partie là se mots dans ces amendements du gouvernement et de madame Di Folco, je me serais rangé à cet avis, et j'ai, je l'aurais volontiers voté, même si les les termes de, de, de, de, de départements de France ou de régions de France reste, je préfère les amendements présentés par tous mes collègues et par moi-même.

j'ai réveillé tout le monde, ben oui, mais de temps en temps, il faut bien, donc je vais le défendre Monsieur le Ministre, mes chers collègues, puisque nous avons tous déposé le même : tout d'abord, je crois qu'il est aussi important de le dire, d'abord parce qu'effectivement cette proposition de loi et je crois que nous avons tous sur appelé d'ailleurs avec beaucoup de force et de sincérité des expériences que nous vivons dans nos départements et de la difficulté aussi à être élu local et si aujourd'hui nous sommes un certain nombre d'a déposé le même amendement, ce n'est pas simplement pour faire durer le plaisir, entre guillemets, mais parce que je crois que nous devons en toute humilité, mais nous garder de vouloir opposer telle ou telle et parce qu'en fait, l'agression envers un un édile, quel qu'il soient finalement qu'il soit un élu local, qu'il soit un élu national ou européen est en fait effectivement madame la robe la rapporteure propose une formulation qui, je le pense et je l'espère. En tout cas fera consensus mais avant d'avoir connaissance de cet amendement, nous avons à toutes et tous, puisque il n'y a qu'à voir la multiplicité de ces amendements pour le reconnaître, pu déposer cet amendement, je crois simplement que, et je veux le dire vraiment ce qu'il voudra, explications de vote ici. Faisons attention dans tous les cas, tout d'abord à 2 choses hein l'agression qui peut être fait en direction d'un élu local ne peut pas être source d'interprétation pour qui que ce soit et justifier as l'existence de telle ou telle structure et nous devons demeurer vigilants deuxièmement parce que je viens de l'entendre, je crois, faisons aussi attention le débat politique a parfois ses forces et ses faiblesses, et donc ne renvoyons pas tout devant la justice ce qui relève du débat contradictoire et parfois de la virulence du débat démocratique. Merci, cher collègue, et enfin le l'amendement. Numéro 18 Madame avait, il est défendu, madame la présidente merci, cher collègue. L'amendement numéro 6 présentée par Madame Goulet. En réalité, Monsieur le Ministre, ma la présidente l'amendement va dans le même sens : il s'agissait évidemment d'élargir le dispositif, je crois que c'est fait, il est défendu. Merci l'amendement numéro 13 Monsieur Bénard Roche. Oui, le président abondement en fait a pour objet d'inclure l'outrage sexiste, inscrit à l'article 621 du code pénal dans la liste des agressions et des violences commises sur les élus pour être des droits à la constitution de partie civile, les associations nationales d'élus, les réflexions sur le physique, les suspicions d'illégitimité, les commentaires et de liées au genre je bascule mais par exemple, a dit : j'ai été à à la réunion de tous les Verts de la région PACA pour signer le contrat territorialisation de la planification écologique entre la ministre, la première ministre et et le président de la région sans monter sur scène 19 élus pour signer le contrat 17 hommes et de femmes donc octobre quand on dit tout ça est réglé dans tout ça n'est pas réglé voilà donc je reprends le sexisme perdurent en politique, il est important d'offrir toutes les garanties de protection aux femmes politiques qui subissent des agressions, le réseau élues locales élus ES a notamment révélé en 2021, que plus de 74 % des femmes élues locales subissent des comportements et des remarques sexistes dans le cadre de l'exercice de leur mandat, le cyber sexisme des femmes en politique est également être augmentation exposées à des formes de violence amplifié en Ligue en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle, ces violences dissuade souvent des fables de s'engager durablement politique pour ces raisons, il est nécessaire d'aider les femmes élues qui souhaite engager des procédures judiciaires pour être accompagnés par des associations nationales d'élus tout au long de leur parcours judiciaire et même si vous me direz que c'est Andorre, je pense qu'il est utile de mentionner clairement l'outrage sexiste. Merci, cher collègue, et nous allons maintenant passer à l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements, madame la rapporteure. Oui, madame la présidente, merci mon avis sera assez rapide puisque, évidemment, un avis favorable à un moment du gouvernement qui est identique, autre puisque c'est une une coproduction fructueuse ensuite concernant les autres amendements qui sont par le même que les autres mais il a la même finalité, donc c'est un avis défavorable puisque il est satisfait avec l'amendement du gouvernement et le mien est identique pour les amendements suivants, les amendements 5 rectifier bis 7 rectifié bis, 9 10 11 12 14 16 et 18, donc ce sont des demandes de retrait puisque ils sont satisfaits par nos amendements et concernant l'amendement de Monsieur Bénard Roche qui est donc différent puisque il il pointe l'outrage sexiste, le choix qui a été fait par notre amendement et de ne pas faire une liste des infractions pour être le plus large et le plus clair possible donc l'inclusion nominale d'une infraction ne nous paraît pas souhaitable, pourquoi parler de outrage sexiste et pas d'autres outrage qui pourrait exister l'outrage qui figurent dans la proposition de loi est au sens très large, donc c'est une demande de retrait sinon un avis défavorable. Merci madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, sur ces amendements, Madame la Ministre, pardon. Merci madame la présidente, moi je voudrais dire d'abord aux sénateurs, je voudrais saluer leur esprit de responsabilité et les synergies qu'il y a eu entre le Sénat et le gouvernement sur l'amendement de Madame la rapporteure et du gouvernement, ils sont identiques et rédigé de concert, donc vous pouvez comprend que, évidemment, nous y sommes favorables concernant l'amendement du président, la mention monsieur le Président de mentionnant l'AMF ne crée pas de rupture d'égalité, d'autant plus qu'elle figurait déjà dans l'article de depuis l'insertion de cette disposition dans le code de procédure pénale, par la loi du du 15 juin 2000, donc notre critère de décision étant l'efficacité est-ce que oui ou non l'AMRF pourra venir en soutien des élus victimes en se constituant partie civile à leurs côtés, la réponse est oui, et donc je vous propose un retrait au profit des amendements qui ont été validé l'amendement du gouvernement et l'amendement de la rapporteure pareil concernant les dix amendements identiques, je partage bien sûr la volonté de certains d'entre vous d'étendre la possibilité de se constituer partie civile, mais là aussi, ces amendements, puisqu'ils ont été satisfaits par les deux premiers amendements et sur l'amendement du Monsieur le Sénateur Bénard Roche je vous propose aussi le retrait de cet amendement au profit de ce que nous avons déposée. Merci madame la ministre, alors il y a une demande d'explication de vote de madame De Lattre. De souligner simplement qu'il n'y avait pas d'opposition sur l'ensemble des associations d'élus, mais simplement de ma part le fait de, de saluer les associations, l'association des maires de France, association des départements de France et régions de France, qui ont travaillé avec moi depuis le début sur cette proposition de loi nous avons travaillé avec madame la rapporteure et le gouvernement sur l'amélioration de cette PPL, c'est tout le sens de nos niches et du travail que nous pouvons faire en profondeur dans ces commissions ce travail de coconstruction avec le gouvernement et l'élégance qui a eu madame le rapporteur de me demander mon avis avant de défendre de déposer cet amendement pour savoir si en tant que auteur de cette proposition de loi, j'étais d'accord, bien évidemment, je suis d'accord avec toutes les améliorations que nous avons porté ensemble, tous ensemble, ici sur les bancs du Sénat et j'espère qu'ils seront portés de la même force et même conviction sur les bancs de l'Assemblée nationale, parce que, encore une fois, au nom de l'efficacité de la loi et pour que justice soit rendue à nos élus, merci à vous en tout cas moi je vous invite à voter les amendements de la rapporteure et du gouvernement. Il vous

petite originalité dans ces amendements, à savoir que le texte madame De Lattre s'adresser d'abord à la protection des élus locaux, nous sommes bien d'accord avec cela et je me suis pas trompé, sauf erreur, et dans un 4ème alinéa de l'amendement madame Di Folco l'extension, donc de cette protection est étendue aux membres du Sénat de l'Assemblée nationale et du Parlement européen. Si vous voulez être efficace mais chers collègues n'oubliez peut être pas aussi les membres élus de la 3ème, chambre de la République, le seize. Et pourquoi, enfin, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas élus, ils sont quand même dans une chambre d'et vous avez aussi d'autres membres qui sont ceux de du Conseil de l'Europe, ce sont des élus qui sont, qui siège au Conseil de l'Europe, donc très honnêtement étendre à d'autres chambres que l'objectif initial qui était celui de défendre les élus locaux, voilà peut créer éventuellement des interrogations que je tenais quand même à partager avec. Merci, cher collègue, la parole est à madame Vogel. Merci madame la présidente, je viens en défense de l'amendement numéro 13, mon collègue Guy Bénard Roche pardonnez-moi pour la violence des propos qui viennent et ils ne sont pas de moi, ils sont juste adressé à moi, c'est ce que je reçois quotidiennement sur les réseaux, grosse pute, pute Walk retournent à la cuisine connasse retournes sucer de l'enturbanné connasse islamo-gaucho connaissent de laïcards de Lesbos c'est assez équilibré, quand même, as un problème avec la religion chrétienne, ferme ta gueule écologiste de merde, les gens comme toi, vous êtes cuit vos têtes seront sur des piquets manges merde que tuer tu là où tu manges bon ça j'ai jamais compris les gens comme moi, n'attendent qu'une chose : le signal pour faire la peau aux gens comme toi, vous avez sans doute eu envie de me couper, madame la présidente, et je vous comprends, c'est inacceptable, et comme toutes et tous, ici, je considère ces propos intolérables, pourtant ce n'est qu'un infime, infime échantillon des insultes et des menaces que je reçois quotidiennement, notamment sur les réseaux sociaux et je suis très loin d'être la seule parce que oui, quand on est une femme en politique aujourd'hui, on se fait harceler dès qu'on existe un peu exagérément, selon certains, dans l'espace public et c'est un problème démocratique, parce que c'est cela mène de nombreuses femmes à s'autocensurer à disparaître des réseaux sociaux par peur pour leur vie ou pour se protéger, mentalement et ça pose un problème démocratique parce que les femmes élues qui sont déjà minoritaire partout sont moins visibles et audibles à cause de ces violences et j'entends très bien que, juridiquement, vous considériez que l'inscription de l'outrage envers un ou une élue soit suffisant mais comme vous l'avez entendu ça tout trajets spécifiques, tant par sa violence, sa fréquence et par sa nature même le fruit de la domination patriarcale, voilà pourquoi je vous demande de voter d'abord l'amendement porté par le groupe écologiste afin d'inclure les spécificités de l'outrage sexiste dans la liste des agressions et violences dont vous entendez protéger des élus dans ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Wattebled. Bien, la parole est à monsieur Laménie. Oui merci madame la présidente, madame la Ministre, monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, alors je me rallie re-bien entendu la vie de la madame le rapporteur de la commission des lois, donc je l'amendement 7 rectifié bis de notre collègue, Madame Noël et plusieurs de nos collègues, collègues, mais je dirai quelques mots sur l'amendement de Monsieur Ben, qu'on peut comprendre bon l'actualité égalité femmes-hommes et pour les mômes qui font partie de la délégation égalité femmes-hommes au sein du du Sénat, bon, c'est aussi des sujets réellement d'actualité qu'on peut partager, même si il y a quand même eu une évolution je dirais dans dans les conseils municipaux, les conseillers départementaux, conseils régionaux, la place des femmes est importante et on peut le dire aussi au Sénat il y a des collègues, sénatrice de très grande qualité donc je je tiens, je le dis sincèrement, hein, je le dis sincèrement voilà donc je crois il y a quand même eu une évolution positive positive même si je dirais on n'a pas complètement encore l'égalité, bon voilà, il faut le dire, donc, alors donc je voulais me rallier vraiment et et puis aussi que salué l'initiative de notre collègue Nathalie Delattre et puis ce ce travail de grande concertation qui a été fait et je crois que c'est des sujets parce que beaucoup critiquent les élus à tout niveau, ben il parle sans savoir, bien souvent, et lève toutes les formes d'agressivité, de violence, comme cela a été largement souligné et je crois que c'est un combat permanent, un combat collectif qui mérite réellement respect, reconnaissance, voilà merci.

je me suis je vais être casser l'ambiance mais je vais l'assumer parce que je crois que vous voyez, à un moment donné à toujours vouloir détailler et faire des liste à la Prévert, on en arrive dans nos propres excès que pour autant nous voulons contrôler empêcher et moi j'entends et vraiment mais je j'ai compris, je partage l'indignation, ma chère collègue de ce que vous venez de nous lire. Mais je pense que cela effectivement relève, à un moment donné, d'une attaque personnelle à l'égard d'une. Sénatrice et donc il y a là 2 solutions : le combat politique. Et donc nous allons au combat et quand nous allons combattre. Donnons des coups et nous acceptons nous recevoir, où effectivement ce que vous pouvez juger comme une attaque personnelle et qui est justifié au nom de l'exercice du mandat et donc il faut pouvoir porter plainte, mais ça ne peut pas être l'un ou l'autre en permanence culpabilisant compte et on va se le dire très tranquillement comme ça nous arrange nos accusateurs et on se Servent comme ça nous arrange aussi, ce qui nous chantent des louanges parce que oui c'est difficile aujourd'hui de faire de la politique dans une société qui est fracturé dans une société où la violence n'a jamais été aussi forte et donc à un moment donné, nous sommes les catalyseurs inévitablement de cette violence et je m'excuse, je m'en emporte et parce que je crois que c'est un moment donné, des choses que nous vivons toutes et tous, nous avons tous autant que nous sommes ici ce soir, un rapport différents réseaux sociaux parce que nous gérons différemment la violence qui peut exercer et ce que moi je peux ressentir peu pour un autre ici, être un non événement. Parce que ce que vous dites et violent, mais parce que moi je pourrais vous raconter aussi mon histoire et je pense avoir plus souffert en arrivant ici, d'avoir été une jeune sénatrice plus que d'être une femme, sénatrice, mais parce que ça, c'est la ville chacune et de chacun et donc à un moment donné, sachant garder raison quand il y a, attaques d'un élu personnel oui, la justice et la et les associations d'élus doivent être au rendez-vous, si nous pensons que c'est du ressort du chant et du combat politique, la reine démocratique nous est ouverte affrontons nous menons les combats qui sont les nôtres et sachant ne jamais renoncer à nos idéaux.

Madame la présidente, madame la Ministre, monsieur le ministre, monsieur le président, madame le rapporteur, je trouve que notre débat est extrêmement important est extrêmement important parce que nous sommes partis grâce à Nathalie Delattre, que je remercie sur ce sujet qui nous a déjà fort occupé dans la loi Engagement et proximité, qui est l'attaque physique d'élus dans l'exercice ordinaire de leurs fonctions ordinaires qui est de porter la voix de de la loi et, aujourd'hui naturellement nous évoque aussi un certain nombre d'autres violences qui pèse sur des élus, moi je félicite Cécile que Carmen pour son intervention, elle était pleine de passion, mais elle était très juste, je pense qu'ici les uns et les autres, nous avons au travers des réseaux sociaux des listes de compliments et ne de mots insupportable comme ce que vous avez évoquée chers collègues dans d'autres registres, et qui ne sont pas acceptables, mais je pense, et Cécile Cukierman a raison, je pense qu'il nous faut rester sur un sujet qui est celui d'où nous parlons avec le mot d'outrage qui couvre l'outrage sexiste mais aussi l'outrage raciale, moi j'aimerais aussi qu'on parle tout autant de celui-là et que je pense qu'on est en générique Catherine Di Folco elle apporter une réponse dans laquelle je crois, chacun peut se retrouver et ensuite il y a le combat politique et des plaintes qui peuvent être déposée pour diffamation contre nous, comme nous pouvons en déposer, donc cher collègue, moi je compatis à ce que vous dites, encore une fois, si on pouvait échanger tous les commentaires qu'on a sur nos réseaux, je pense qu'il y aura un florilège de plaisanterie de très mauvais goût et haineuse, mais les choses sont ainsi et je pense que cela relève plus de la dérive des réseaux sociaux plutôt que d'autres choses et j'un dernier mot pour monsieur Cannet cher Patrick Kanner, moi j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour vous, mais alors là je suis en total désaccord avec vous l'émission de Monsieur Hanouna. Je regrette même de prononcer son nom, mais il existe, il fait des émissions, j'ai regardé l'émission dont vous parlez, le début, hé ben moi j'ai pas la même analyse que vous, je veux dire quand on est provocateur et qu'on va chercher les coups, on ramasse des coups, y compris des coûts qui sont pas pardonnable et qui sont maladroits et je ne pense pas qu'on puisse comparer ce qui s'est passé dans cette émission avec ce que le maire de signes ou d'autres ont vécu leur faire contre nature. Merci.

les dispositions de cette proposition de loi aux 3 collectivités du Pacifique par compte et pour ma parfaite compréhension le troisièmement de votre amendement madame la rapporteure et monsieur le ministre, vous avez voulu préciser l'assemblée de Corse pour les élus régionaux territoriaux et de l'Assemblée de Corse, vous m'a pas fait de compréhension quid, les élus de l'assemblée de Polynésie française, les élus du Congrès de Nouvelle-Calédonie et les élus de l'assemblée territoriale de Wallis et pour Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre, peut être, vous voulez répondre. Sur ce seul point parce que c'est point je je. Attends madame la sénatrice d'inquiétude légitimes, les élus sont compris dans le texte, on n'a pas oublié d'élus donc, soyez rassurés, la déclinaison que vous avez fait d'élus qui ne sont pas des métropolitains, naturellement, nous les avons pris en considération dans le texte, bien sûr, bien sûr, il y a aucune exclusion sur les absolument rassurer. Madame la rapporteure veut compléter peut être. Oui, pardon, en fait, si le rajout a été fait sur la suggestion de de régions de France, parce que justement il fallait spécifié l'assemblée de Corse, qui est une spécificité, voilà qui ne se retrouvent pas dans région de France et il fallait préciser les élus territoriaux justement pour préciser vos territoires.

voilà madame la rapporteure, donc nous précise que la formulation qui était présenté couvre bien les territoires, en tout cas de la Polynésie, c'est ce que j'ai compris. Il n'y avait plus d'autres demandes d'explications de vote. Donc avant de procéder au vote des 2 amendements identiques de madame le rapporteur et une Monsieur le Ministre. Au nom du gouvernement, je voudrais m'assurer des amendements qui ont été retirés Monsieur Kader vous le maintenez.

donc voilà je vous remercie. Et donc je mets aux voix nos deux amendements 19 et 20. 3 identique madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, qui est pour.

qui est contre qui s'abstient, il est adopté, après l'article. 1er nous avons le 3 rectifier, il est présenté par Monsieur Merci à madame la présidente, madame et monsieur les ministres, nous avons tous partager le constat suivant : lors de la discussion générale, le phénomène de violence à l'égard des élus grandit hélas trop bien connu des maires et des personnels municipaux, ceux-ci se retrouvent souvent seuls à devoir faire face d'une part, un nombre grandissant d'infractions et d'autre part à des agressions, menaces, intimidations, insultes, injures qui les touchent dans l'exercice où, du fait de leur fonction mais qui touche également les membres de leur famille auprès offrir une réponse à cela, j'avais déposé une proposition de loi visant à lutter contre les incivilités menaces et violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, elle avait pour objet de renforcer la réponse pénale en cas d'agression d'élus ou de dépositaire de l'autorité publique, les amendements donc je que je dépose vise à compléter la proposition de loi notre collègue Nathalie Delattre. Ce premier amendement fait référence à l'article 85 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles une personne peut se constituer partie civile, nous proposons d'y ajouter une dérogation en précisant que les conditions de recevabilité d'une constitution de partie civile, notamment le délai de 3 mois ne s'applique pas aux personnes dépositaires de l'autorité publique, cette nouvelle disposition permettra aux victimes d'ouvrir une instruction sans tarder, je vous remercie. Merci madame la présidente, alors cet amendement tend à prévoir que les agressions contre les élus pourront permettre la constitution immédiate de parties civiles, je rappelle que pour toutes les victimes, cette constitution n'est possible qu'en cas de refus d'engager des poursuites ou après 3 mois, les exceptions sont déjà prévues, notamment pour les crimes et pour les infractions commises lors des élections, il ne paraît pas nécessaire d'aller au-delà, au risque de faire des élus, des victimes, à part ce n'est pas du tout la volonté en tout cas de l'auteur de la proposition, la commission des lois, donc, a émis un avis défavorable. Merci madame la rapporteure, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Oui pour le gouvernement En réalité, oui, il ne s'agit pas de faire des élus une catégorie particulière mais par ailleurs. Je comprends parfaitement le sens de votre amendement. Vous pensez être peut être plus efficace, mais en même temps on va perdre de la réactivité de la rapidité, je rappelle, je le fais tout à l'heure dans le discours, on peut en reparler, mais un certain nombre de, de, de, de directives ont été données pour que très rapidement on traite toutes les infractions qui concernent les élus. Mettre en branle immédiatement l'instruction par le truchement d'une plainte avec constitution de partie civile c'est y ajouter de la lourdeur et je pense que on va perdre le bénéfice d'une enquête qui est parfois ultra-rapide si vous avez des constatations immédiates à faire dans le cadre de l'infraction flagrante, on peut les faire en quelques en quelques heures si le parquet est saisi, il les diligences, ça va très très vite, si vous allez vous constituer partie civile, il va falloir qu'il y ait une consignation, il va falloir que l'on désigne le juge d'instruction et vous prenez également le risque d'une disparition de la preuve, donc je comprends parfaitement le sens de votre amendement très franchement, il ne me semble pas sur le terrain, dans les principes, je vous suis sur le terrain, il ne me paraît pas aller vers ce vers quoi vous souhaitez c'est-à-dire une répression peut être plus plus plus rapide en tous les cas, si c'est de la rapidité, on va la perdre si c'est de la fluidité, on va perdre au sein, on a un risque de dépérissement de la preuve et je vous invite monsieur le sénateur tout en partageant l'objectif qui est le vôtre et qui est le nôtre d'ailleurs et je pense que nous l'avons tous démontré en travaillant je vous incite l'impératif naturellement mais est interdit lorsque je m'adresse à vous retirer votre amendement, sinon c'est une position évidemment de Roger. Merci, monsieur le Ministre, Monsieur Gold. Non, j'ai bien entendu les arguments, on va retirer l'amendement. Je vous remercie l'amendement 3 rectifier et retirer les nous avons un amendement de rectifier toujours présenté par Monsieur goal. Oui, madame la présidente, je pense que dans le même esprit que l'amendement précédent donc certainement avec les mêmes avis il s'agit de nuancer le principe de l'aménagement des peines en s'assurant qu'en cas de jugement aboutissant à une peine d'emprisonnement le juge puisse prononcer un mandat de dépôt qu'on se Coupable, même s'il fait appel afin que la peine s'applique sans délai. Si Madame la rapporteure. Oui, madame la présidente, cet amendement pose plusieurs questions mais il paraît satisfait dans l'esprit par l'article 397 tiré quatre du code de procédure pénale et par ailleurs, il revient sur le principe de l'aménagement des peines de moins d'un an, ce qui ne paraît pas du tout souhaitable, donc la commission a émis un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. des concepts qui ne vont pas ensemble des principes qui ne vont pas ensemble, donc, là encore, je comprends parfaitement le sens de votre amendement alors on on va dire les choses, le tribunal correctionnel peut décerner un mandat de dépôt contre le prévenu qui comparaît libre s'il prononce une peine d'emprisonnement d'au moins un an ou en cas de récidive, quelle que soit la durée de l'appel, voilà les textes et s'il prononce une peine d'au moins 6 mois, il peut décerner un mandat de dépôt à effet différé, je pense que aller au-delà serait déraisonnable et comme la raison et notre boussole dans le cadre de l'examen de ce texte de la même façon que précédemment, je vous propose un retrait sinon le gouvernement se verra dans l'obligation de vous dire, monsieur le sénateur qu'il est défavorable à l'amendement que vous avez déposé. Merci, monsieur le Ministre, il est donc retiré. Et nous passons au hein rectifier Monsieur Gold. Toujours dans dans le même esprit, madame la présidente, ce dernier amendement a pour objet de prévoir une traduction du prévenu sur le Champ en cas d'infraction commise sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou sur un membre de sa famille, je ne vois pas dans ce cas de figure, ce qui justifie que le parquet dispose d'une marge de manoeuvre, d'autant que le garde des Sceaux a fait par la circulaire du 7 septembre 2020 de la nécessité d'une réponse pénale systématique et rapide, alors pourquoi ne pas le faire dans la loi ce que permettrait mon amendement. Merci madame la rapporteure. en l'état du droit, il s'agit effectivement d'une faculté pour le procureur l'amendement monsieur Gold 2, rendrait la comparution immédiate obligatoire mais l'appréciation portée par Kurer nous semble importante pour la qualité des poursuites cet amendement pourraient dès lors nuire à la qualité de la réponse pénale et vous venez de le dire Monsieur Gold, vous souhaitez qu'il ait une réponse rapide et pour ce faire, nous pensons que la réponse se trouve dans l'application de la circulaire du garde des Sceaux, que vous avez vous-même ciné signalé et qui demande effectivement procureur d'agir systématiquement et rapidement, donc c'est un avis défavorable. Merci madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, même avis. Oui du lutter contre ma modestie naturelle ce sénateur, je pense que la circulaire est largement suffisante érigée en principe, bien sûr, on comprend là encore le sens de l'amendement, il faut aller vite, il ne faut pas perdre de temps, il faut une réponse immédiate, efficace, c'est notre voeu commun, de là à contraindre par un texte, le procureur de la République à ne plus avoir de choix, ça me paraît excessif, donc Monsieur le sénateur, je vous demande là encore de retirer votre amendement, faute de quoi je me verrai dans la tristesse de vous dire que le gouvernement il est défavorable. Non.

On vous donnera la parole à l'amendement suivant éventuellement alors. En avril. Nous allons passer à la présentation par Madame la rapporteure de l'amendement numéro 20. Oui, rapidement, il s'agit de supprimer l'article de puisque tout le dispositif a été intégré à l'article 1. D'ailleurs, Monsieur le Ministre. Merci si Monsieur Boyer veut avec retardement prendre la parole, on va lui proposer de le faire maintenant. Je vous remercie, madame la présidente, je voudrais revenir sur les amendements qui ont été déposés par mon collègue Éric Gold je comprends tout à fait le la la démarche qui est la sienne, je comprends aussi la réponse qui est faite, mais on a trop de cas, on a beaucoup trop de cas où effectivement la réponse qui est faite vis-à-vis des agresseurs n'est pas assez rapide, on a des exemples dans notre département ou dans d'autres départements où on a des eu des agressions sur des élus ou la réponse qui a été fait, vers les agresseurs, a dû a traîné pendant 6 mois,

des consignes qui soit donnée au procureur pour que les choses puissent s'accélérer et aille plus vite, on a eu dernièrement une réunion de l'association des maires dans notre département où, effectivement, beaucoup d'élus, pas mal d'élus se sont plaints de la Länder des de la lenteur des procédures qu'il y avait vis-à-vis des agressions contre les élus, et je crois que il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là, en dehors des procédures qui, il y a en on peut, on peut parfaitement le comprendre, mais que je pense qu'il faut que les choses aillent beaucoup plus vite, on s'aperçoit que des fois, dans certaines situations, je ne dirais pas vers qui il dans quelle situation les choses vont beaucoup beaucoup plus vite.

Il s'abstient, il est adopté, et donc l'article 2 est supprimé. à l'article 3 un amendement 22 présentée par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, c'est un amendement de coordination dans un, dans Très bien, merci madame le rapporteur favorable je mets aux voix l'amendement 22 avec l'avis favorable de la commission. Qui est pour, qui contre qui s'abstient, il est adopté, je mets aux voix, l'article 3 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté, nous avons un amendement 21 il est présenté par Madame la rapport. Alors c'est aussi un amendement de coordination, puisqu'il s'agit de changer le type de la proposition de loi pour la mettre le mettre en adéquation avec la réécriture du texte. merci Monsieur le Ministre. De ce que le Sénat, le gouvernement Madame la rapporteure, madame la présidente, de nous avions travaillé ensemble sur ce texte. Et je pense qu'on a raison de le faire, je constate également qu'au-delà des divergences politiques politiciennes, il y a des sujets qui sont transpartisan, je m'en félicite également, je voudrais ajouter une toute petite chose au-delà de notre volonté commune d'aller de l'avant, j'ai pris un certain nombre de mesures, je les ai rappelé tout à l'heure, mais je voudrais vous rappeler que parmi les contractuels, que l'on a envoyé dans toutes les juridictions, beaucoup de procureurs ont souhaité dédier un contractuel aux élus. Certains ont créé une ligne téléphonique dédiée, une boîte Mail dédiée. C'est contractuel dédié, parfois c'est un substitut parfois, c'est le procureur lui-même se rende auprès des élus, j'avais été extrêmement frappé de constater que un jeune élu dans la région de Dijon ne savait pas ce qu'était pour un maire que de venir que de devenir pardon, officier de police judiciaire et donc ces réunions, elles se font et ça marche plutôt pas mal, parce que les magistrats du parquet sont très investis dans ses missions que j'ai souhaité renforcer pour autant, pour autant, il y a, comme on le dit avec cette métaphore sportive quelques trous dans la dans la raquette et de temps en temps, on vient me dire mais nous. On n'a jamais rencontré le procureur on le le contractuel dédié, on sait pas qui c'est, bon j'ai un exemple très précis en tête, c'est le maire d'une petite commune dirai pas laquelle, qui a accepté sur son territoire, la construction d'un établissement pénitentiaire, dites-moi, c'est pas rien quand on sait les réticences parfois de le compatriote avoir ce type d'établissement s'implanter et je lui dis : des cours d'une visite et d'un café qu'ils m'offrent très gentiment dans sa mairie, mais vous avez rencontré le procureur, elle me dit : non, je ne sais pas qui c'est, donc là, moi il m'est interdit de donner, vous le savez, des directives individuelles au procureur, hein, je le dis à certains l'oublient parfois et, en revanche, je peux rappeler les termes d'une circulaire comminatoire, alors je voulais vous dire que souvent au cul agir les uns et les autres vous venez me dire, mais telle mère de mon territoire, à des difficultés, voilà et n'hésitez pas à le faire parce que la chancellerie est ouverte aux élus bien sûr, je suis moins proche que vous des maires, évidemment, mais certains maires viennent me racontait cela, il faut le prendre en considération, bien sûr, et le régler, comment on fait. C'est pas très compliqué, on dit au procureur général, monsieur le procureur général, je vous rappelle les termes de ma circulaire veiller à ce qu'elle soit mise en oeuvre, c'est pas plus compliqué que ça, d'ailleurs au prochain salon qui va se tenir dans les jours qui viennent, salon des élus, il y aura, pour la première fois un stand justice en face du stand du ministère de l'Intérieur, mais symboliquement, c'est extrêmement important, voilà ce que je voulais vous dire il y a ce que l'on fait dans le cadre de l'évolution normative et puis il y a des bonnes pratiques et moi je peux vous assurer que les magistrats du parquet sont très investis auprès des élus, parfois il y a quelques hésitations, on va le dire comme ça de façon leucémique pour ne heurter personne quelques tergiversations oui voilà et donc là, le garde des Sceaux et c'est son rôle, intervient pour dire : attention aux élus, il faut les soigner comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont la République. Merci, monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement présenté par Madame la rapporteure au nom de la commission des lois qui un avis favorable du gouvernement. Manque qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il était adopté, et je mets donc on voit l'intituler ainsi modifié, qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il être adopté, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Il y a-t-il des demandes d'explications de vote. Alors nous commençons par Madame. Un petit mot juste pour remercier une dernière fois l'ensemble de mes collègues qui ont participé à à cette à cette rédaction ce compromis Madame la rapporteure merci Chère Catherine, Madame la Ministre, Monsieur le garde des Sceaux, merci encore une fois, pour ce travail, co-construit comme l'on dit très constructif et vous demandez effectivement de pouvoir parrainer ce texte auprès de l'Assemblée nationale, nous le ferons, porté par nos élus députés mais nous comptons sur vous pour porter cette parole, celle du Sénat, auprès de l'Assemblée nationale et faire en sorte que ce texte passe très rapidement et qu'ils puissent pouvoir effectivement rentrer dans la loi et est rentré en fonction, le plus vite possible parce que, encore une fois, les élus le réclame depuis longtemps et c'est juste rendre justice merci.

cette présenté cette loi, on trouvera bien une niche quelconque pour la la allez suivre le processus parlementaire, comptez sur nous. Merci madame la ministre, avant de passer la parole à Madame Gatel vous dire que vous pouvez vous préparer à un scrutin public pendant les explications de vote, donc Madame Gatel vous avez la parole. Merci madame la présidente, nous vivons l'été rappelé par beaucoup de collègues dans une société nerveuse et agressive ou toute personne porteuse d'une autorité peut être un moment agressé, il en est ainsi des élus et, comme chacun, j'ai une pensée particulière pour les élus locaux, encore une fois, je remercie Nathalie Delattre et ses collègues pour nous permettent d'aller au-delà de ce que nous avons fait d'engagement et proximité et permettez-moi de me souvenir de ce jour où nous avons appris le décès du du maire de signer le choc violent qui a été le nôtre de réaliser soudainement qu'un élu pouvait mourir parce que un jour ordinaire il exercer sa mission et je voudrais monsieur le garde des Sceaux, vous rendre hommage parce que suite à à la loi Engagement et proximité, il y a eu un silence il y a eu aussi un changement de gouvernement, enfin bref ce qui est important, c'est voter la loi, mais aussi s'assurer de son suivi, il se trouve qu'à l'époque, je vous ai écrit au nom de la délégation pour savoir ce que devenait tout ce que nous avions voté et vous avez répondu en adressant des circulaires au procureur et considérant que les sénateurs pouvaient continuer à s'intéresser aux choses qu'ils avaient fait je vous avez invité à la délégation aux collectivités pour venir présenter le bilan de ce que vous avez fait, cher collègue, moi, je vous invite à demander au garde des Sceaux pour chacun de vos départements, ce qui a été fait, puisqu'il a fourni une fiche pour chacun des collègues, des membres de la délégation et je salue ce qui se passera en terme de de rendu de justice après une agression, mais je voudrais aussi souligner tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire le fait qu'il y a aujourd'hui, dans beaucoup de territoires un dialogue normal et naturel entre un procureur et les maires, alors que certains ignoraient les autres et les autres et parfois peur des procureurs, ensuite, vous avez parlé de tous les moyens que vous avez mis à disposition de la mobilisation qu'il y a aussi de la part des associations d'élus en terme de formation et je pense qu'aujourd'hui c'est terrible et tragique, mais les élus doivent être préparés à vivre des situations difficiles et à se retrouver dans des situations d'agression Ford, merci encore une fois aux collègues pour cette proposition de loi, merci monsieur le garde des Sceaux et continue à nous fournir des fiches de suivi, c'est extrêmement. Si bon coup merci madame Gad Madame Goulet. mais un le président de la le ministre monsieur le garde des Sceaux évidemment remercier Nathalie Delattre et et constater les progrès accomplis depuis 2018, 2019 depuis les tragédies dont on vient de parler après le rapport de Philippe Bas après la loi, engagement de proximité après aussi vos engagements, Monsieur le Ministre, que viennent rappeler Françoise Gatel tout ça est un travail sur la durée qui concerne ne les élus, on ne réglera pas tous ces problèmes sans évidemment travailler sur la violence et la délinquance, en règle générale et les incivilités, il y a aussi tout un travail de prévention, les élus sont vraiment de proximité dans dans nos territoires, nous y sommes évidemment très attachés, et je crois que ce qui s'est passé ce soir, dans cet hémicycle, est de nature à les rassurer sur l'accompagnement à la fois des parlementaires, mais aussi du gouvernement pour la poursuite sereine du mandat qu'ils exercent et nous on dont nous avons évidemment besoin puisque c'est eux qui qui assurent le maillage de la France et évidemment la représentation comme au long dit du premier échelon de la démocratie, donc je crois qu'on a fait du très bon travail depuis toutes ces années, entre le travail de Françoise Gatel les les travaux, vous avez conduit vous-même les travaux de de Philippe bah évidemment, je crois que tout ça est extrêmement utile à un exercice serein d'une mission qui est indispensable à la République. Merci, cher collègue Monsieur Wattebled. Merci ma main présidente monsieur le garde des Sceaux, monsieur, la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, chacun connaît l'adage, nécessité fait loi et malheureusement cette proposition de loi s'avère nécessaire, je tiens donc à remercier notre collègue Delattre auteur de ce texte, ainsi que le groupe RDSE pour l'avoir inscrit dans leur niche réservée je tiens également à celui d'avancer, de la Commission, ouvrant la possibilité pour l'assemblée parlementaire, le Parlement européen et l'école qui territoriale de se porter partie civile en cas d'agression d'un de leurs membres ou de ses proches, face à ce fléau intolérable, chacun doit pouvoir prendre sa part les chiffres ahurissants de cette recrudescence à la violence à l'endroit des élus ont été rappelés pour l'écrasante majorité ce sont des élus agressés, maire adjoint, ils sont en première ligne face au déchaînement de colère de certains de leurs concitoyens leur courage et leur pneus pugnacité tout à chacun au respect. Puisque le sentiment d'impunité contribue à augmenter les violences verbales et physiques, la question des les instructions et la traduction des prévenus et centrale face à ces violences, les s'inquiète et appréhende d'appliquer leurs pouvoirs de police, avec le peu de moyens dont il dispose, a une autre devoir de soutenir pleinement en cas d'agression, d'agression, mais également au quotidien, avant que le pire ne se produise, c'est pourquoi, avec mon collègue du Nord Jean-Pierre le col, nous avons proposé depuis plusieurs mois dans tous les arrondissements, le département des réunions aux élus locaux, afin de leur donner les moyens pour pouvoir réagir face aux inciter et au comportement violent, ces réunions sont organisées en compte en coopération avec les sièges préfectoraux les procureurs de la République, les gendarmeries et les commissariats aussi pour toutes ces raisons, ou c'est très bien que le groupe indépendant voudra en faveur de ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur.

le plus beau des textes, la plus belle des lois ne produira pas ses effets, si on ne donne pas, on avons, nous avons nous le Sénat avec le gouvernement travailler de concert pour obtenir ce résultat, autant maintenant il appartient au gouvernement de poursuivre, vous disiez tout à l'heure monsieur le garde des Sceaux, qu'un maire du secteur de Dijon ne connaissait pas le procureur, je peux vous dire que je connais beaucoup moins des maires de leur département qui ne connaissent pas le procureur, je veux dire par là que des procureurs sont souvent très occupé et n'ont pas le temps d'aller en direction des des maires, moi, je forme le voeu que demain il sera différemment et que les procureurs et les maires pour se parler plus souvent merci à notre présidente. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Bénard Roche. Merci madame la présidente, bien sûr, qu'une loi telle que celle-ci, une proposition de loi pour soutenir les édiles victime d'agression est nécessaire, utile et salutaire. dire le contraire c'est se voiler la face, dans une société qui devient de plus en plus violentes et où, en fait, tout ce qui contribue à la bienveillance et au respect des être s'humains, quels qu'ils soient devient. Un peu, comment dire. Aléatoire ou surprenant ou stupéfiants à tous les niveaux, qu'il s'agisse des élus qu'il s'agisse d'autres personnes, qu'il s'agisse des fois de l'accueil des migrants ou d'autres problèmes qui peuvent se poser à nous sommes dans une société qui vit de cette façon-là, en particulier par les réseaux sociaux, nous l'avons évoqué et donc toute avancée qui permettrait de venir en aide aux gens qui sont victimes de violences et d'agressions ne peut être que salutaire, j'ai, j'ai fait part de nos réserves, qui porte sur cette sorte d'ultra spécialisation de la justice qui consisterait à adapter les règles en fonction des victimes ou d'une catégorie de victimes

pour autant, bien entendu, nous comprenons très bien qu'il faille. Protéger les, les, les, les élus et les représentants de la nation et que donc il s'avère nécessaire de pouvoir les aider dans leurs démarches, en leur permettant effectivement ce que permis ce texte voilà donc, c'est pour cette raison-là et parce que nous, nous souhaitons que ce vote soit fait à l'unanimité que nous voterons bien entendu cette proposition de loi et et que je me permettre dernière réserve je, je l'ai dit,

Terminé du rues d'accord très bien. Alors je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé proposition de loi visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus, de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agressions. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe RDSE sur la proposition de loi, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Alors, voici donc le résultat. Du scrutin alors sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence 32 votants, 300 quarante-quatre nombre de suffrages exprimés 344 pour l'adoption 344, le Sénat a adopté à l'unanimité. L'ordre L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération. à la suite d'une décision de cour d'assises, présenté par monsieur Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues demande du groupe Rassemblement démocratique et social européen. Hein, monsieur le président, vous avez la parole. Merci madame la présidente, madame et monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, je le dis ça ne dis tour cette proposition de loi à tout un texte arrive strictement juridique et procédurale et qui ne soulèvera sûrement pas les foules, seulement elle lui la réparer un rouage non négligeable de notre institution judiciaire puisqu'il est question de modifier l'article 377 du code de procédure pénale afin de clarifier les conditions dans lesquelles l'arrêt rendu par la cour d'assises peut valoir titre de détention en effet cet article a fait leur billet d'une réécriture il y a un an suite à la loi du 22 décembre 2001 2000 maintient pour la confiance de l'institution judiciaire et puis qui et plus spécifiquement dans un article 6 qui comportait diverses dispositions relatives à la cour d'assises, parmi ces dispositions, l'une d'entre elles a eu pour objet d'abandonner l'exigence pour la Cour de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de l'accusé ayant comparu libres lorsque celui-ci était condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans cette loi a prévu que si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle, l'arrêt de la cour d'assises vos dit de de détention sans qu'il faille est décerné un mandat de dépôt spécialement motivée et pour obtenir ces résultats, il a fallu réécrire l'article 367 du code de procédure pénale, en toute transparence, sa tactique est difficile à lire, et il y a encore plus pour celui qui n'est pas juriste, pourtant c'est dans sa réécriture que se trouve le noeud du problème, aussi je vais m'efforcer d'être plus athlétique possible, voilà ce que prévoit la rédaction actuelle cet article. d'abord, une personne condamnée à une autre peine que la prison n'est évidemment pas incarcéré tout comme une personne condamnée à une peine de prison déjà couverte par la durée de sa détention provisoire d'ailleurs cas une personne condamnée à plus de 10 ans de prison, c'est-à-dire la réclusion criminelle qu'elles soient détenus au long au moment de la décision se verra immédiatement incarcéré à la suite du juge Halphen 3ème cas une personne condamnée à moins de 10 hommes de prison si elle n'est pas détenu au moment du jugement, on pourra se voir délivrer un mandat de dépôt directement par la cour d'assises et ainsi être incarcéré dès le jour du jour, voici les 3 seuls cas visés par le texte, or il y a un gars qui a été oublié, celui d'une personne détenue au jour du jugement et condamné à une peine de prison de moins de 10 à un détail qui aura échappé aux députés, aux sénateurs, aux membres du gouvernement et à l'ensemble de nos collaborateurs et comme redouté que je ne lis pas chaque matin les revues d'actualité Judy juridique, le droit pénal, c'est finalement L article d'un journal satirique paraissant le mercredi, que le général de Gaulle, appelé le volatile, à savoir le canard gêné du 27 avril 2022 qui m'aura mis la puce à l'oreille, seulement, quelle est la conséquence d'une telle oublie le légiste et il dit qu'elle peut être radical, à savoir la libération d'un condamné malgré la condamnation à une peine de détention

portant application de l'article 367 du code de procédure pénale, ce décret règle la difficulté en autorisant expressément la cour d'assises a délivré un mandat de dépôt lorsqu'il personne est condamnée à moins de 10 ans quelle que soit sa situation au jour de la condamnation, seulement je n'a pas de moi à personne ici la teneur de l'article 34 de leur constitution la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables la procédure pénale : l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats,

la détermination des conditions dans lesquelles l'arrêt rendu par la cour d'assises pas vouloir de détention relève donc du domaine législatif si, comme le groupe B RDSE que la lettre la Constitution sans respecter je vous proposerai d'adopter cette proposition de loi que notre rapporteur Maryse Carrère améliorer en simplifiant encore davantage la rédaction pour que notre droit soit lisible et efficace, mais avant de juger la parole, j'aimerais dire un dernier mot sur la cause réelle et profonde de cette proposition de loi, outre les questions de mandat de dépôt de comparution et de réclusion criminelle, l'autre sujet cette PPL et celui de l'inflation législative et la surcharge du calendrier parlementaire, nous dit souvent que dans cet hémicycle, combien il est de plus en plus difficile de bien écrire la loi les procédures accélérées donc plus rien exceptionnelle pour le prendre qu'un exemple, qui se souvient encore que le délai normal entre l'examen en commission et la gamine Serge public n'est pas d'une semelle, comme si à chaque fois le cas désormais mais bien deux semaines

mais c'est aussi la conséquence d'une tendance qui, jusqu'au mois de juin dernier était particulièrement flagrante, nous examinons trop de textes déjà que trop long dans l'élite, trop court, c'est aussi de cela dont il est question de cette proposition de loi, j'espère que nous adopterons

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par le président Jean-Claude Requier et plusieurs membres du groupe RDSE porte sur un sujet assez technique, puisqu'elle concerne les règles d'incarcération d'un accusé condamné par la cour d'assises, tant que l'arrêt n'est pas définitif, dans l'attente d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, cette proposition de loi vise plus plus plus précisément à corriger une malfaçon législative figurant à l'article 367 du code de procédure pénale, dans un souci de sécurité juridique cette malfaçon s'est produite à l'occasion de l'examen de l'année dernière, du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté comme rédactionnelle qui est à l'origine de la difficulté que je vais vous exposer dans un instant, lors de l'examen du texte au Sénat, nous n'avons pas bien mesuré la portée de cet amendement, qui était passée relativement inaperçue au milieu de dispositions plus que contenait le projet de loi depuis 2011, l'article 367 du code de procédure pénale prévoit que l'arrêt de la cour d'assises condamnant l'accusé à une peine privative de liberté vos titres de détention si les condamné l'accusé et donc incarcéré à l'issue de l'audience sans qu'il soit nécessaire de décerner un mandat de dépôt à moins bien sûr que la durée de la peine soit déjà couverte par la détention provisoire, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a voulu assouplir le principe selon lequel l'arrêt de la cour d'assises vos titres de détention afin de tenir compte de la situation des personnes qui comparaissent libres devant la cour d'assises et qui, et qui ne sont finalement condamné qu'à une peine correctionnelle pour ces personnes, une incarcération systématique à l'issue de l'audience n'apparaît pas forcément nécessaire dans cette hypothèse, la loi dans prévu que l'incarcération ne serait plus automatique et elle a laissé le soin à la cour d'assises de décerner un mandat de dépôt, si elle estime que les éléments du dossier, justifie une mesure dans l'hypothèse où l'accusé comparaît détenu, il était en revanche envisager de maintenir le principe selon lequel la au titre de détention si l'accusé a été placé en détention provisoire, il paraît en effet logique de l'incarcérer à l'issue de l'audience, s'il est condamné à une peine privative de liberté le problème provient de la modification introduite à l'Assemblée nationale qui a restreint l'application de ce principe à l'hypothèse d'une condamnation à une peine de réclusion criminelle, plus rien n'est prévu en revanche dans le cas où l'accusé qui comparaissait détenu et condamné à une prennent de peines d'emprisonnement de nature correctionnelle, c'est-à-dire à une peine inférieure à 10 ans d'emprisonnement une lecture littérale de l'article 367 du code de procédure pénale pourrait conduire à libérer l'accusé qui était jusqu'ici placé en détention provisoire, alors qu'ils viennent d'être condamné à une peine de prison ferme, une telle solution ne serait pas cohérente et elle n'est pas conforme à l'intention du législateur d'après les informations que j'ai recueillis au cours de mes auditions cette malfaçon législative n'a pas entraîné à ce jour de conséquences fâcheuses aucune libération inopportune n'est à déplorer et aucun contentieux n'a été recensé, qui aurait été comme qui aurait le 25 février dernier, le gouvernement a pris un décret qui a clarifier les règles applicables en rappelant que l'accusé qui est détenu au moment où l'arrêt rendu, et qui est condamné à une peine d'emprisonnement ferme doit être incarcéré cette disposition est cependant fragile juridiquement puisque la procédure pénale relève après un principe du domaine de la loi, c'est la raison pour laquelle je vous invite à adopter la proposition de loi que nous examinons ce soir, en espérant qu'elle sera inscrite rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, je signale pour terminer que la commission des lois a adopté avec un accord avec l'auteur de la proposition de loi 2 amendements, le 1er à procéder à une réécriture du texte afin d'en proposer une réalise une rédaction plus concise, les auteurs de la proposition de loi s'était inspiré de la rédaction du décret qui énumère de manière très pédagogique, toutes les hypothèses pouvant être rencontrés, il nous a semblé préférable d'apporter une correction plus ponctuelles afin d'éviter que la loi soit redondantes avec le décret le 2ème amendement concerne l'application outre-mer sous des dehors très technique, le texte poursuit donc vous le vous l'avez compris un objectif très concret, puisqu'il s'agit d'éviter que des personnes condamnées potentiellement dangereuses soit remise en liberté de manière intempestive, je ne doute pas qu'il recevra pour cette raison un large sourire soutiennent sur tous les bancs de notre assemblée. Je vous remercie, Madame la présidente. C'est le président de la commission des lois, monsieur le Président, Ruquier. Madame la rapporteure Carrère, mesdames et messieurs les sénateurs, la procédure de jugement des crimes par la cour d'assises présente, nous le savons tous une importance toute particulière, à raison de la gravité des faits pour lesquels la Cour de se prononcer, mais également en raison des conséquences de cette décision pour les justiciables qui le souhaitent, accusée ou victime cette procédure doit donc être aussi satisfaisante et et, juste que possible. C'est la raison pour laquelle la la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire que j'ai eu l'honneur de porter dans une véritable co-construction avec le Sénat. Et votre commission des lois, monsieur le président, buffet à modifier en profondeur les règles relatives au jugement des crimes par la cour d'assises, l'objectif était de les rendre plus cohérentes d'assouplir les modalités de composition de la cour d'assises. De simplifier le déroulement des audiences de renforcer le rôle du jury populaire et d'accroître les possibilités d'individualisation des sanctions prononcées. Par ma profession. Mon expérience et mes convictions, vous savez, je suis extrêmement attaché au respect de la souveraineté populaire du jury, c'est également grâce à cette loi, que le président de la cour d'assises à l'occasion de son rapport introductif à l'ouverture des débats, expose désormais les éléments à charge et à décharge, tels qu'il résulte de l'information et non tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, c'est enfin grâce à cette loi qui ont été modifiées les règles relatives à l'incarcération à l'audience de l'accusé, condamné prévue par l'article 367 du code de procédure pénale afin de renforcer l'individualisation des décisions rendues par la cour auparavant l'incarcération d'une personne qui comparaissait libre et tête automatique, y compris lorsqu'elle était condamné à une peine d'emprisonnement, c'est-à-dire à une peine inférieure à 10 années. D'emprisonnement, et alors même que l'accusé pouvait faire appel de la décision, ou on appelle formé un pourvoi en cassation désormais si l'accusé est libre au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement par exemple à une peine d'un ou 2 ans, la cour doit, par décision spéciale et motivée, décider, ou non, et c'est là tout l'intérêt de cette évolution de décerner un mandat de dépôt, la cour doit donc se pencher spécifiquement sur la question de savoir si l'incarcération automatique de l'accusé, alors qu'il comparaît libre à l'audience, laquelle se tient souvent plusieurs années après les faits, est nécessaire si, par exemple, c'est un exemple, l'accusé a respecté à la lettre. Son contrôle judiciaire. Cette évolution renforce l'oeuvre de justice en permettant à la cour d'apprécier au cas par cas, si l'incarcération immédiate du condamné est nécessaire si elle permet de le sanctionner à sa juste hauteur si elle permet de favoriser sa réinsertion car je le rappelle, la peine doit évidemment et impérativement répondre à ces objectifs. Toutefois. à la suite de modifications apportées lors de la discussion parlementaire le texte définitivement adopté comportait une ambiguïté puisqu'il ne traitait pas de la question des accusés détenus condamnés pour Crime ou délit à une peine d'emprisonnement. J'ai complété. La partie réglementaire du code de procédure pénale par un décret du 25 février 2022, qui est venu lever cette ambiguïté, en indiquant que, pour les accusés détenus, il n'était pas nécessaire de décerner un titre de détention ainsi si l'accusé comparaissant détenu devant la cour, et condamné à une peine d'emprisonnement, l'arrêt de la cour d'assises vos de détention. Bien évidemment, il est également pertinent que cette ambiguïté soit levée par la loi, comme le prévoit le présent texte du président Ruquier. Qui avait, je le supposé été alerté sur cette problématique par des praticiens de la cour d'assises et qui en réalité a lu un hebdomadaire que nous sommes très nombreux à lire. L'article unique de cette proposition de loi modifie ainsi l'article 367 du code de procédure pénale afin de clarifier l'hypothèse de l'accusé détenu condamné à une peine d'emprisonnement par la cour d'assises pour prévoir que ce dernier doit évidemment rester détenu après sa condamnation, c'est d'ailleurs l'esprit du texte, le gouvernement est d'accord avec l'évolution normative que vous proposez, je tiens donc à remercier chaleureusement le président Ruquier pour sa vigilance et l'ensemble de son groupe pour conclure je tiens également à saluer le travail d'amélioration rédactionnelles menée par Madame, la rapporteure Carrère sur cette disposition qui permet d'aboutir à un texte plus concis et de davantage mettre en valeur la modification apportée. Merci, monsieur le Ministre, dans la suite. De la discussion générale, la parole est à monsieur Jean Roux pour le groupe RDSE.

Madame la présidente, monsieur le ministre madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, j'aimerais avant tout saluer la vigilance aiguë dans ta et fait preuve le président Jean-Claude Requier sur un sujet qui, malgré sa technicité est d'une importance particulière. Je ne vais pas entrer à mon tour d'un trop de détails et de complexité, tout a déjà été dit de ce point de vue avec une grande virtuosité juridique tant par l'auteur de la proposition de loi que par notre rapporteur Maryse Carrère, la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a de modifier l'article 367 du code de procédure pénale ainsi à la R fait évoluer une nouvelle fois les conditions d'incarcération ou de libération des personnes jugées par la cour d'assises, et plus particulièrement les conditions dans lesquelles l'arrêt rendu par la cour d'assises peut valoir titre de détention au cours de cette réécriture, il a été décelé un oubli rédactionnelle aux conséquences potentiellement grave, nous rappelant que la procédure pénale n'est pas une affaire technocratique cet oubli concerne le cas où une personne jugée par une cour d'ASUS et déjà en détention et est condamné à une peine d'UTA 100 inférieur à 10 ans il est en effet nécessaire de reformuler une partie de l'article 367 du code de procédure pénale afin que la cour d'assises, puis se par décision spéciale et motivée, décidé de décerner mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu lors du prononcé de l'arrêt et condamné pour Crime à une peine d'emprisonnement ferme, mais sans pour autant que la peine prononcée, constitue une peine de réclusion criminelle, je salue la rédaction adoptée par notre commission des lois, qui poursuit l'esprit du texte initial, tout en lui offrant plus de simplicité, de lisibilité, cette solution s'inspire du décret du 25 février 2022, que le gouvernement avait adopté afin de ne pas de pallier ce vide législatif, comme ça a pu être souligné, il est à craindre que ce dispositif actuellement en vigueur soit frappée d'inconstitutionnalité puisqu'ils ne respectent pas la répartition des domaines de compétence entre le législateur et le pouvoir réglementaire prévues aux articles 34 et 37 de notre constitution, heureusement, à ce jour, personne n'a encore fait de recours Direct ou contre le décret mais nous ne saurions laisser notre droit dans un tel état de rue karité et très naturellement le groupe RDSE sera favorable au dispositif législatif proposé, il a parlé donc essentiel que ce texte arrive au terme de la navette parlementaire durant ces prochaines semaines pour éviter toute déconvenue, enfin, pour faire écho aux propos introductif du type du président Ruquier je voudrais à mon tour souligner que nous sommes face ici à une des conséquences de l'encombrement du calendrier parlementaire, les lois sont trop nombreuses, trop longue, parfois bavarde et d'ortho Loire dans dans le rythme parlementaire nous conduit à mal travaillé sur des dispositifs certes techniques mais non sans implication concrète les conditions qui ont mené à l'émergence de ce texte illustré hélas trop bien les conséquences de cette méthode, cela me rappelle, dans un autre genre, les propositions de loi répété sur l'élection des juges consulaires sur ce sujet aussi, le Sénat a été vigile hein, grâce notamment à la mobilisation de notre collègue Nathalie Goulet a conclusion, vous l'aurez compris le groupe RDSE votera sans réserve cette proposition de loi. Merci monsieur Roux, la parole est à Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la reporter, mes chers collègues. Si la loi n'a pas tous les droits comme le rappeler, Mireille Delmas-Marty, elle possède néanmoins une utilité et une place certaine au sein du droit comme l'article 34 de la Constitution, le consacre le droit a besoin de la loi et, surtout, d'une voix claire intelligible et réfléchi, le réalisateur a donc une grande responsabilité, celle de faire de bonnes lois, c'est aussi l'objet notre discussion aujourd'hui la proposition de loi présentée par le président, Ruquier et 12 de nos collègues complète des dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération, suite à la décision d'une cour d'assises, cette proposition de loi surtout, corrige une malfaçon introduite à l'Assemblée nationale dans la loi dite confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2020 T1 pardon dont nous étions rapporteur avec mon collègue Philippe Bonnecarrère en effet, cette loi n'avait pas prévu le cas où un accusé détenu devant la cour d'assises et condamné à une peine inférieure à la réclusion criminelle, soit moins de 10 ans d'emprisonnement à ce moment-là la Cour pouvez décerné un mandat de dépôt afin de pouvoir l'incarcérer immédiatement cette omission dans la loi signifier qu'un condamné pouvait être remis en liberté, immédiatement après le rendu du du jugement, une situation que le ministère de la Justice a cherché à résoudre en comblant cette carence par le décret du 27 février 2022 : une solution temporaire, mais très fragile, si l'on peut se lever cette tentative réglementaire, seule une disposition législative permettait, selon l'article 34 de remplir cet oubli, lui seul pouvait jeter des bases solides et apporter une solution pérenne pour résoudre c'est là cette lacune ah si la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui reprend l'esprit du décret évoquer avec néanmoins une recherche de simplification poussée par une rédaction concise et claire en effet la rapporteur de la commission des lois, madame pardon attendu à clarifier au mieux le texte afin de le rendre plus accessible ainsi la proposition de loi modifie le code de procédure pénale si nous pouvons nous féliciter de résoudre une fois pour toutes et par la bonne voie législative cette carence regrettable, il est nécessaire de nous interroger tout de même sur les raisons qui nous amènent à nous réunir, une fois de plus, à une heure tardive pour combler un trou dans la raquette, produite par des lois établies souvent dans la précipitation, cette urgence ne permet pas d'apprécier les conséquences réelles des mesures adoptées grâce notamment à une véritable étude d'impact préalable c'est seulement lors de leur implication effective qu'apparaissent alors ces erreurs législatives l'inadéquation avec la pratique et tout aussi souvent du nous le savons, à un enchevêtre ment complexe de ces règles, la justice pénale est aujourd'hui en France une parfaite illustration depuis plusieurs années, nous déplorons ici au Sénat la complexification des lois des codes et procédures l'inflation normative et législatives car lorsque la loi devient bavarde les l'essentiel disparaît souvent au profit de l'accessoire, la superposition des textes juridiques sans aucune refonte globale contribue elle aussi à l'opacité des règles,

peu praticable en effet entre 2008 et 2022 le nombre des articles du code de procédure pénale législatif est passé de 1522 à 2403 je formule le voeu aujourd'hui que nous puissions engager cette réforme essentielle de la procédure pénale, cette réforme, qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, je rappelle les délais de jugement des crimes atteignent toujours près de 50, moi mon groupe votera donc cette utile, proposition de loi du président Ruquier largement améliorée par la rapporteure Maryse Carrère. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre. Jean verse laine pour le groupe, les indépendants. Madame la présidente, monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission madame le rapporteur, mes chers collègues, en 2021 sur 32000 affaires suivies par des juges d'instruction 700 arrêts ont été prononcées par les cours d'assises à la suite d'un procès, ce qui représente environ 2800 auteur mise en accusation. Les affaires portées devant la cour d'assises ne représente qu'une part minoritaire de la totalité des affaires pénales, toutefois, elle concerne les infractions les plus graves de notre droit, la procédure relative à ses affaires se doit lors d'être irréprochable. La proposition que nous examinons aujourd'hui porte sur des dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale qui règle le sort de l'accusé, une fois que la cour d'assises, a rendu son arrêt. Par souci de simplification, une loi de 2011 prévoyaient que l'arrêt de la cour d'assises, titre de détention sans qu'elle n'ait besoin de décerner mandat de dépôt. Souhaitant apporter plus de nuances à ce principe, la loi du 22 décembre dernier a sans le vouloir laisser subsister un vide juridique sur les hypothèses dans lesquelles l'arrêt de la cour d'assises vos titres de détention. En effet, un qu'a été omis, celui où l'accusé détenu au moment où l'arrêt rendu, et condamné à une peine inférieure à 10 ans d'emprisonnement heureusement cette situation, ça a été dit, ne s'est jamais présenté. C'est pourquoi, pour éviter les délibérations inopportune, le décret du vingt-cinq février dernier à remédier à cet oubli. Cependant, selon l'article 34 de la Constitution, les règles de procédures pénales doivent être fixées par la loi la proposition de loi reprend alors toutes les hypothèses visés dans ce décret, cette initiative est en effet essentiel à plusieurs égards, déjà parce que la loi pénale doit être précise et prévisible, chacun doit savoir à quoi ils s'exposent et dans quelles conditions et ensuite dans une démocratie. Le lien entre la société et la justice, je veux dire le lien de confiance, il était indispensable, et pour les victimes, mais aussi pour les citoyens, il serait inconcevable de remettre en liberté un détenu condamné à une peine d'emprisonnement, même de façon temporaire, en raison de lacunes rédactionnelle ou législatives en outre la rédaction simplifiée de la commission apparaît tout à fait complémentaires aux dispositions du décret de l'exécutif enfin appliquer ces mesures en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie dans les îles Wallis et Futuna, semble totalement légitime, avant de conclure : je tiens à saluer la qualité des travaux de la rapporteure Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité territoires.

Madame la présidente, monsieur l'auteur que je remercie à l'époque de la concentration des médias, de continuer à soutenir la presse indépendante en la lisant. Madame la rapporteure, que je remercie énormément pour la clarté de vos explications qui a éclairé éclairer notre regard sur ce point sur ce point très important et particulier monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, voilà devant un texte qui n'a en fait d'un ou dès que la simplicité de son objectif, mais relève et révèle plusieurs points cruciaux de notre système, il s'agit, disons-le clairement, comme l'a rappelé, notre rapporteur de corriger une malfaçon législative enfer est pavé de bonnes intentions, on peut aussi dire que il ne faut pas confondre vitesse et précipitation sur des adages trop souvent répétée, mais qui trouve pourtant encore dans notre processus décisionnel la loi pour la confiance de l'institution judiciaire a voulu mettre en oeuvre des recommandations d'un rapport de 2008, préconisant une simplification des modalités d'incarcération libération suite au prononcé de l'arrêt des cours d'assises. Vous connaissez ma méfiance je suis pas le seul d'ailleurs envers le terme de simplification qui parfois dans les modifications apportées à notre système pénal sa campagne par exemple ici d'une mise à l'écart de juges là d'une baisse du niveau des droits de la défense mais idée ici ne peut et n'a pu que faire l'unanimité et peut s'exprimer d'une manière certes la décision de la Cour vos titres de détention pour les cours d'assises et les tribunaux correctionnels la possibilité de voir cette décision comme nécessaire et suffisante pour l'incarcération de justifiables condamné a subi une erreur rédactionnelle, vous l'avez parfaitement expliqué en limitant cette faculté en cas de condamnation criminelle, elle en correctionnelle si la gestion de cette erreur qui peut être un peu problématique puisque erare Oumanou Metz tu persévères arrêt diabolicum l'erreur et Tibet devait persévérer dans son erreur est plus problématique et devant cette difficulté que nous venons de révéler le gouvernement a publié un décret correctif à décret bé comment oser croire que ce gouvernement, monsieur le garde des Sceaux est entendu clarifier la situation, par un simple décret, vous, vous nous l'avez expliqué mais un des fondements de notre société et que les règles de droit pénal sont fixées par la loi et par les représentants du peuple j'dit que cela relève de notre société, mais toute l'acceptabilité du droit pénal et de sa procédure trouve racine dans une loi votée par ses pairs, puis par le fait d'être jugé par ses pairs, via des jurés populaires dans les cours d'assises, ce qui peut être mis à Bâle avec la généralisation à venir des cours criminelles départementales dont le rapport vient de vous être remis par le comité, qui comprend des parlementaires dont Maryse Carrère et moi-même, alors je sais que ce président et ses gouvernements successifs sont friands de légiférer par ordonnances et leur multiplication inquiétant d'ailleurs fait l'objet d'un suivi justifier pendant 30 mais la procédure pénale, elle relève bien dans l'article 34 de la constitution du domaine de la loi, je profite de ce moment pour encourager le gouvernement a concentré enfin d'actions dans la publication des décrets d'nécessaires à la bonne application de la loi, quelle que soit la loi qui était votée par le Parlement, aussi, pour ce qui est de ce texte afin d'éviter tout recours pour contester d'incarcération au motif d'absence de base légale, le groupe RDSE, que je remercie dans sa liste, le texte que nous, alors je pense de manière unanime, voter afin de réparer l'erreur initiale du texte de loi par Bluetooth réunis et l'erreur de tentative de réparation inadapté par décret prise là pas le gouvernement, notre groupe d'votera pour ce texte. Merci monsieur la parole est à monsieur Thani Mohamed Soihili pour le groupe RDPI. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux sur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, vous l'avez rappelé cher président Ruquier l'objectif de cette proposition de loi de loi et simple, mais pour autant essentielle puisqu'elle vient corriger de malfaçon issu de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, ceci n'avait rétabli l'obligation pour la cour d'assises de décerner mandat de dépôt à effet immédiat ou différé que lorsque l'accusé comparaissait libre et qu'il était condamné à une peine d'emprisonnement ferme, laissant un vide s'agissant des détenus comparaissant détenus un décret du 25 février 2022 portant application de l'article 367 du code de procédure pénale pallier cette incongruité afin d'éviter que certains accusés ne soit remis en liberté par les juridictions en prévoyant le cas dans lequel l'accusé comparaissait détenu et était condamné à une peine d'emprisonnement ferme, la commission des lois a, par la voix de ses rapporteurs madame Maryse Carrère retenu une rédaction plus concise pour préciser que l'arrêt vaudra titre de détention lorsque l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises, ces dispositions seront également étendu à Wallis et Futuna, hein, Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le groupe RDPI ou votera donc la proposition de loi ainsi modifiée l'examen de ce texte de montre une nouvelle fois que le législateur n'est pas infaillible, je suis moi-même intervenu il y a tout juste un mois, en tant que rapporteur d'une proposition de loi visant à réparer de malfaçon législative introduite par la loi, pacte en 2019 lors de la réforme du régime électoral des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, ce n'est finalement qu'une illustration supplémentaire des limites de la procédure accélérée et de notre propension à légiférer dans l'urgence, elle-même induite par la densité de nos travaux, compte tenu de l'heure du jour chargé du Parlement, peut-être serait-il opportun d'envisager de regrouper au sein d'un seul et même texte les corrections, comme celle-ci, enfin, et nonobstant cette malfaçon législative qu'renfermé, je tenais à profiter de mon temps de parole pour souligner rapidement, rassurez-vous, les avancées de la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire, je pense notamment au procès filmé aux enquêtes préliminaires limité à 2 ans au secret professionnel des avocats ou encore à la généralisation des cours criminelles au 1er janvier 2023 qui sont à l'expérimentation dans 15 départements depuis septembre 2019 je suis conscient de la réticence de certains concernant cette dernière mesure est moi même très attaché à la persistance des jurés populaires qui sont l'expression de la participation des citoyens à la justice mais je tenais à rappeler que les réformes des cours des cours d'assises ont toujours été réalisé avec parcimonie en 20 ans, c'est la quatrième, que l'on connaît et que la mise en place de ces cours. A déjà permis l'abaissement du taux d'appel, la réduction du délai d'audiencement et d'éviter que certains crimes sexuels ne soient correction n'Alizée, un autre les jurés populaires subsisteront au sein des cours d'assises traditionnelles pour toutes les infractions punies de plus de 20 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'un appel, si l'on se réfère aux crédits alloués à la justice, ces 3 dernières années, je ne vous ferai pas offense monsieur le garde des Sceaux en vous disant que sans moyens, un magistrat, un personnel judiciaire pour mener ces audiences géants locaux pour les accueillir, d'heure utilité sera relative sinon nul. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président. Madame la présidente, monsieur le Ministre, je le garde des sceaux, madame la rapporteure, Monsieur, président de la commission des lois, mes chers collègues, merci, comme mes autres collègues à Jean-Claude Requier pour cette proposition de loi qui a repéré que ce soit par un canard déchaîné ou un conseil juridique, peu importe, mais en tout cas, il a repéré un dysfonctionnement qui nous a contraints à une torsion de notre système durant plusieurs mois en effet, sur un plan constitutionnel effectivement et ça été rappelé par tous nos collègues. La détermination des peines relève du domaine de la loi article 34 le règlement sorti que 37, or dans le cas précis qui nous occupe aujourd'hui, il n'y a pas de dispositions législatives suffisante actuellement le le cas d'un accusé déjà détenu condamné à une peine d'emprisonnement, donc par définition, une peine qui ne peut que c'est les dix ans est réglé par décret manière je dirais aléatoire sur un plan constitutionnel cette solution palliative ne fait que masquer un défaut et n'existe que pour éviter que certains mandat de dépôt de soit privée de fondement légal qui est d'ailleurs prévu de reprendre dans la loi le dispositif existant, prévu dans le décret par le décret du 25 février 2022 pris par vos soins, monsieur le garde des Sceaux, l'objet de la discussion n'est donc pas le fond, mais mes chers collègues, la forme, car on ne saurait se satisfaire de cette situation qui ne respecte pas les dispositions, donc de notre constitution, en l'espèce, cette situation qu'on ne peut que regretter nous contraint aujourd'hui à avoir un débat. Qui n'en est pas hein, puisque sur le banc, aujourd'hui, personne ne remet en cause la nécessité de respecter la répartition du domaine législatif est du domaine réglementaire en effet privé une personne d'une liberté publique, en l'occurrence la liberté d'aller et venir, ne peut relever que le domaine de la loi, n'en déplaise peut-être incertain le pouvoir réglementaire à un domaine et heureusement circonscrits, tout ne peut pas se régler par voie d'ordonnance et le décret je profite toutefois de cette occasion pour vous faire part d'un sentiment évoqué par d'autres collègues, quant à la fabrique de la loi, le vide juridique qui nous occupe aujourd'hui a été crée par les modifications apportées au code de procédure pénale, par la loi de 2021 dans pour la confiance dans l'institution judiciaire lors de nos débats de l'époque, nous n'avons pas remarqué cette situation et il est vrai qu'à relève d'un oubli. On peut gloser sur si c'est un manque de temps ou autre chose en tout cas ce manque de temps est à mes yeux, surtout due à une pratique qui est devenue la norme, cela fait maintenant plusieurs années que l'examen de la majorité des lois par le Parlement se fait par la voix de la procédure accélérée, or cette procédure appelée procédure d'urgence jusqu'en 2008 n'avait vocation, comme son nom l'indiquer à être utilisé qu'exceptionnellement, en cas d'urgence, le fait qu'elle devienne une procédure accélérée est révélateur de l'objectif poursuivi durant le quinquennat son créateur, monsieur Sarkozy, son utilisation n'était plus lié à l'urgence, mais à la volonté d'écourter les débats sa banalisation participe de l'affaiblissement du Parlement puisqu'elle abrège la discussion parlementaire, cette pratique a d'ailleurs pu être utilisé par des gouvernements auxquels j'ai aussi appartenu. Mea culpa, Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République en a même fait un argument de campagne en 2017, je cite, je cite, la procédure accélérée devra être la procédure par défaut de l'examen des lois afin d'accélérer le travail législatif. Cette promesse de campagne a été manifestement tenu pourtant tout juste intronisé, fort d'une majorité de soutien très large, à l'Assemblée nationale à l'époque et disposant de tous les instruments du parlementarisme rationalisé pour mener à bien ses réformes, Emmanuel Macron, président de la République n'avait pas besoin d'accélérer le temps de délibération parlementaire, on le voit aujourd'hui le temps d'examen nous a manqué en l'espèce, et si j'étais un peu cynique ou facétieux, je dirais que nous devons aujourd'hui prendre du temps à examiner une proposition de loi qui ne fait que corriger un manque de temps, alors prenons le temps de la réflexion, mes chers collègues, interrogeons-nous sur la manière dont nous souhaitons finalement travailler ne confondons pas l'urgence d'une situation et l'empressement de nos gouvernants car in fine, et c'est la qualité de nos travaux qui en pâtissent. Comme le disait non pas le poète mais le professeur de droit constitutionnel Guy Carcassonne que beaucoup d'entre nous ont pu connaître il disait pour faire de bonnes lois, on n'a pas encore inventé mieux que le Parlement. à condition bien sûr de lui laisser le temps de travailler, vous l'aurez compris mes chers collègues, et en remercions nouveau monsieur le Président requis, elle nous souscrivons au rétablissement, prévu dans cette proposition de loi et le groupe socialiste à l'unanimité, votera en sa faveur. Merci monsieur le président, la parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe CRCE. Si madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous me permettrez, avec le respect que j'ai tout d'abord pour le groupe RDSE et leur proposition de loi, le respect pour chacune et chacun en train de ramasser mon propos et donc inévitablement d'aller à l'ascension à l'essentiel, sans être forcément caricatural, tout d'abord pour rappeler que la précision apportée par la PPL visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération à la décision d'une cour d'assises est intéressante puisqu'effectivement, mais ça a déjà été rappelé par nombre des intervenants avant moi, elle permet de clarifier les dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance en institution judiciaire était sur ce point, lacunaires et je n'ouvre pas ici le débat de comment devons-nous faire la loi pour qu'elle soit la meilleure possible, je rappellerai cependant qu'à l'époque, le groupe CRCE, s'étaient opposés à la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et, bien que nous puissions envisager la pertinence d'un mandat de dépôt dans les cas les plus graves, tels que ceux relevant de la cour d'assises il nous semble que notre groupe se doit d'être cohérent, c'est pourquoi, au vu de notre opposition à la loi relative à la confiance dans l'institution judiciaire en 2021 de notre peau de notre positionnement également contre la surpopulation carcérale, tels que le témoigne la PPL déposée par notre collègue la présidente Assassi visant notamment à mettre fin à cette surpopulation qui elle a pu déposer au mois de septembre 2022, nous nous abstiendrons sur sa proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre madame la rapporteure, chers collègues, le Parlement, votée en 2011 : la simplification des modalités d'incarcération des accusés jugés par la cour d'assises, la condamnation à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subies pouvait alors valoir titre de détention de l'accusé en 2020, le Parlement s'est à nouveau penché sur cette question, le législateur a introduit une exception dans l'hypothèse où l'accusé comparaît libre était condamné à une peine correctionnelle malheureusement cette modification opérée à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a introduit une élève ni rédactionnelle en modifiant les modalités d'incarcération prévue par le code pénal, l'article 367 de ce même code précise que l'arrêt de la cour d'assises pour titre de détention si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle, écartant ainsi l'hypothèse où l'accusé qu'on par les détenus était condamné à une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans la rédaction actuelle de l'article 300 sont 67 entraînerait malheureusement la remise en liberté d'un accusé, placé en détention provisoire avant l'audience, lorsqu'il est condamné à une peine d'emprisonnement ferme, il est donc nécessaire d'adapter notre droit, un décret du gouvernement pris en février dernier a tenté de clarifier les règles applicables à cette situation, précisons chaque cas pour être rencontrés par la cour d'assises, l'arrêt de la cour d'assises, voit ainsi titre de détention si l'accusé par les détenus et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement inférieure à la réclusion criminelle, bien que le décret et probablement parer au plus pressé en tentant de lever l'ambiguïté qui s'était glissée dans l'article 367 du code pénal, les mesures relatives à la procédure pénale, relevons con de lève constitutionnellement du domaine de la loi, ce décret ne pouvait donc régler durablement ce problème de droit, la proposition de loi que nous examinons ce soir enfin ce matin, comporte un article unique, qui nous permet ainsi d'intégrer dans la loi les dispositions prises par le décret du gouvernement, à corriger la malfaçon législative introduite dans l'article 367 du code de procédure pénale lors de la fin, dernier d'efforts, elle précise les mesures applicables lors de l'accusé et condamné par la cour d'assises, non à une peine de réclusion criminelle, mais à une peine d'emprisonnement ferme notre commission des Lois adopté 2 amendements présentés par Madame la rapporteure ajoutant des modifications d'ordre rédactionnel, afin de simplifier la lecture de cet article,

cette redondance et l'allongement de l'article 367 aurait pu prêter à confusion sur les intentions de cette proposition de loi les modifications apportées par la commission permettre une rédaction plus brève afin d'apporter seulement une clarification ponctuels, il est prévu que ces précisions apportées aux dispositions relatives aux modalités d'quand sédation ou de Libération à la suite d'une décision de cour d'assises sont impliqués dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, et de Wallis et Futuna, concerné par le principe de spécialité législative, il était indispensable de corriger rapidement cette et leur pour le bon fonctionnement de nos institutions judiciaires, c'est donc sans surprise que le groupe UC votera cette proposition de loi dans la version amendée pendant tout de commission des lois, je vous remercie. Merci, cher collègue. La discussion générale est Close, nous passons à la discussion du texte de la commission. Je mets aux voix, l'article 1er qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, je mets aux voix, l'article 2 qui est pour. Qui compte qui s'abstient, il est adopté et je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, il y a-t-il des demandes d'explications de vote, il n'y en a pas, je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de Libération à la suite d'une décision de cour d'assises qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient cette proposition de loi est adopté. Mais, chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance, mercredi 16 novembre 2022 à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée.